La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 21 octobre 2021 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la délégation sénatoriale aux entreprises a été publiée. Cette candidature sera ratifiée si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels

Initialement déposée par le député Fabien Matras puis soutenue par le Gouvernement, cette proposition de loi s'inscrit dans la lignée des grandes lois de sécurité civile, au même titre que celle de 1996 relative aux services d'incendie et de secours ou celle de 2004 portant modernisation de la sécurité civile. Avec ce texte, nous avons voulu doter l'ensemble des acteurs de la sécurité civile d'outils modernes et efficaces pour leur permettre d'assurer leurs missions dans les meilleures conditions. Sapeurs-pompiers professionnels, volontaires, marins-pompiers, bénévoles des associations agréées de sécurité civile : je tiens aujourd'hui à leur rendre hommage ainsi qu'à toute la communauté de la sécurité civile, à laquelle j'associe évidemment les personnels administratifs, techniques et spécialisés et les proches des soldats du feu. Devenus également soldats de la santé, ils n'hésitent pas à risquer leur vie pour sauver celle de leur prochain, sur l'ensemble de nos territoires. Sachez-le, mes chers collègues, Patrick Kanner, Loïc Hervé et moi-même avons chèrement défendu les intérêts des acteurs locaux de la sécurité civile tout au long de l'examen de ce texte. Car ils sont, selon nous, le socle de notre modèle de sécurité civile. C'est d'ailleurs sur cette question que se sont focalisés les deux derniers points de divergence demeurant entre l'Assemblée nationale et le Sénat à la veille de la réunion de la commission voire d'obstination, et grâce à l'ouverture d'esprit de nos collègues de l'Assemblée nationale ainsi qu'à notre volonté commune d'aboutir, ces points de divergence ont été surmontés. En ce qui concerne la mise en place d'une expérimentation des plateformes communes de réception des appels d'urgence prévue à l'article 31, nous avions à coeur de conserver les apports

mixte paritaire répond à ces attentes. En effet, le texte prévoit que les conditions matérielles de mise en oeuvre des expérimentations seront définies avec les présidents des conseils d'administration des services d'incendie et de secours et les présidents des conseils de surveillance des établissements de santé concernés. ce qui concerne les carences ambulancières, traitées à l'article 3, le Sénat a toujours considéré que la définition claire prévue à cet article était une véritable avancée, au même titre que la possibilité de différer de refuser les missions relevant de la carence ambulancière afin de préserver les capacités opérationnelles des SDIS. Le Sénat était toutefois attaché à la possibilité de requalifier des missions en carences. Cette précision permettrait aux SDIS d'être justement indemnisés lorsqu'ils ont réalisé une intervention à la demande du 15 dont il s'est avéré par la suite qu'elle relevait en pratique de la carence ambulancière. mixte paritaire répond aujourd'hui à cette préoccupation, puisque l'article 3 conserve la possibilité d'une requalification des carences ambulancières par le si une requête en ce sens est formulée par le SDIS. À la demande des sénateurs membres de la commission mixte paritaire, l'article 3 prévoit également un recours amiable devant une commission de conciliation paritaire en cas de désaccord entre le SDIS et le SAMU. Cette commission paritaire réunira des membres des services d'incendie et de secours et des membres des SAMU afin qu'ils proposent une solution de conciliation dans tous les cas où SDIS et SAMU ne seraient pas d'accord sur le fait que les critères prévus à l'article 3 permettent de qualifier ou non une intervention en carence ambulancière. Nous plaçons beaucoup d'espoir dans la création de cette commission pour apaiser les tensions et réduire le transfert de charges qui existe au détriment des collectivités qui financent les SDIS. Aussi, monsieur le ministre, nous apporterons un soin particulier à l'examen des décrets que le Gouvernement prendra pour donner corps aux commissions paritaires de conciliation ainsi qu'à tous les règlements d'application de ce texte. vous le savez, est rompu à cet exercice. En attendant la publication de ces décrets, mes chers collègues, Patrick Kanner, Loïc Hervé et moi-même vous invitons à adopter sans réserve le texte issu des travaux de la commission mixte

nous pouvons tous être fiers de nos sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, militaires, marins-pompiers, sapeurs-sauveteurs, démineurs, pilotes, mécaniciens opérateurs de bord, bénévoles des associations agréées de sécurité civile, personnels administratifs et techniques des services d'incendie et de secours, mais également des agents de préfecture et des élus de chacun de nos départements qui contribuent chaque jour au secours de nos concitoyens.

madame Dumont, et les membres de la commission mixte paritaire soient remerciés pour leur travail de conciliation. Les équilibres trouvés

chaque fois qu'une catastrophe a frappé le pays les sapeurs-pompiers ont répondu présent : l'ouragan Irma, les inondations dans l'Aude, la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, les pluies dans les Bouches-du-Rhône, l'incendie de Notre-Dame de Paris, les feux de forêt comme cet été dans le Var et dans les Bouches-du-Rhône et les terribles feux de l'été 2017. N'oublions pas non plus leur mobilisation décisive dans la lutte contre la pandémie. Engagés pour tester, mesurer puis organiser la vaccination, les sapeurs-pompiers sont toujours là, prêts à risquer jusqu'à leur vie pour sauver celles des autres.

Cette issue favorable s'inscrit dans l'esprit de consensus qui a présidé à l'élaboration et à l'examen de la proposition de loi, à la fois, à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui ont tous deux adopté le texte à l'unanimité. Je tiens à saluer le caractère équilibré des dispositions qui ressortent de cet accord, auxquelles se sont attachés tout au long de la navette parlementaire les députés et les sénateurs. Cette proposition de loi consacre notre modèle de sécurité civile, notamment au travers de deux dispositions phares que M. le ministre vient de rappeler à l'instant. du rétablissement de la possibilité de requalification des interventions en carence ambulancière, sur la demande du service d'incendie et de secours et par le service d'aide médicale urgente, avec la mise en place d'une procédure contradictoire pour traiter les cas de désaccord potentiels. Je salue plus généralement le fait que le texte donne une définition attendue des carences ambulancières, qui permettra de clarifier le régime des interventions ne relevant pas de la compétence des SDIS, afin que les dépenses ne se rattachant pas à l'exercice de leurs missions ne pèsent pas sur les collectivités territoriales. Cet enjeu sera également traité au niveau des conventions entre SDIS et SAMU, maillons indispensables et complémentaires de la chaîne de secours. Il s'agit, ensuite, de l'expérimentation de plusieurs configurations de regroupement de numéros d'urgence sans supprimer la nécessaire régulation médicale, afin d'aboutir à une solution qui garantisse une plus grande lisibilité et efficacité dans la prise en charge des situations d'urgence. Temps de réponse, qualité d'accompagnement des usagers, prise en charge des victimes, prise d'un premier appel au titre du « débruitage » et bascule vers une plateforme d'envoi des moyens : nous évaluerons méthodiquement au bout de deux ans quelle solution est la plus efficace.

de l'extension de l'accès à la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance, de la prise en charge de la protection sociale par les SDIS ou encore de la facilitation de l'accès au logement social. mesures symboliques, telles que la création d'une nouvelle mention honorifique « mort pour le service de la République » et l'instauration d'un nouveau statut de pupille, ainsi que les garanties apportées en matière de protection des sapeurs-pompiers : durcissement des peines encourues pour outrage à un sapeur-pompier dans l'exercice de sa mission, mission, généralisation de l'usage des caméras individuelles et instauration dans chaque SDIS d'un référent sécurité. Ces dispositions s'ajoutent à la limitation, prévue par un autre véhicule législatif, des réductions de peine accordées en cas d'infraction commise sur un sapeur-pompier. L'amendement de ma collègue Patricia Schillinger, conservé dans le texte de la commission mixte paritaire, permettra de traiter, notamment dans le rapport que le Gouvernement remettra au Parlement, des conditions dans lesquelles le conseil d'administration du SDIS pourrait décider de financer l'allocation de vétérance versée aux sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal. Avec cette commission mixte paritaire conclusive, nous démontrons que l'ensemble des partis républicains soutiennent l'action remarquable de nos pompiers. Il ne pouvait en être autrement lorsque l'on intervient concrètement sur le quotidien de toutes celles et de tous ceux qui font passer la vie des autres avant la leur.

Nous l'avons dit, les attentes sont immenses dans nos territoires pour les acteurs de terrain, professionnels et volontaires, mais aussi pour les associations et les citoyens. Les sapeurs-pompiers sont précieux dans nos territoires et nous ne serons jamais assez reconnaissants à leur égard pour leurs actions et leur engagement quotidien. C'est d'autant plus vrai dans nos territoires ruraux où les sapeurs-pompiers volontaires sont irremplaçables. Il est donc indispensable que les activités de sapeur-pompier volontaire ne soient absolument pas assimilées à celles d'un travailleur, car cela entraînerait la disparition des centres de secours ruraux. Depuis plusieurs années, j'entends les intentions du Gouvernement, qui souhaite maintenir notre système français, lequel donne satisfaction. C'est bien, mais j'insiste : il faut trouver des solutions claires et concrètes à ce problème. Cela doit être une priorité de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, comme vous l'avez indiqué, monsieur le ministre. Plus largement, cette proposition de loi est un véritable texte de consensus. Je me félicite que la commission mixte paritaire soit parvenue à un accord, avec des discussions constructives jusqu'au bout, malgré des points de désaccord finalement surmontés. J'avais ouvert mes propos en première lecture en dénonçant les violences à l'encontre de nos sapeurs-pompiers qui sont en forte hausse. L'article 38 relatif à l'aggravation des peines d'outrage est un début, mais il paraît important de déployer rapidement d'autres outils pour lutter efficacement contre ces agressions inadmissibles. L'expérimentation d'un numéro unique d'appel d'urgence doit nous permettre de construire sur le long terme une plateforme pérenne et efficiente. Néanmoins, il est indispensable que, dans le cas d'appels relatifs à la santé, la gestion de ces appels et les décisions qui en découlent demeurent entre les mains du seul médecin régulateur du SAMU. Cela fait partie

Enfin, une solution de compromis a été trouvée, ce qui marque une avancée. Il faut le dire, les carences ambulancières existent bel et bien,

Je pense notamment à la réserve citoyenne, qui sera très utile, mais également aux dispositions concernant les relations entre employeurs et sapeurs-pompiers volontaires, aux autorisations d'absence pendant

je souhaite rappeler à quel point l'examen de ce texte est un véritable enjeu de société, car il nous invite de nouveau à définir l'ambition que nous assumons pour notre système de secours. La question, somme toute assez simple, est la suivante : sommes-nous prêts à défendre une société de l'engagement volontaire de nos sapeurs-pompiers ? Tous nos concitoyens ont bien conscience que, derrière l'uniforme qui vient les sauver, les secourir, derrière le sapeur-pompier qui est toujours présent quand il le faut, il y a un engagement fort, de chaque instant. Chaque Français peut apprécier les valeurs et les principes qui caractérisent le corps des sapeurs-pompiers. Le volontaire doit être reconnu pour ce qu'il est, c'est-à-dire une personne qui s'engage librement au service de ses concitoyens. On ne peut pas traiter l'engagement volontaire comme on traite n'importe quel autre engagement. Vous le savez, notre système de sécurité civile repose à 80 % sur le volontariat. Il est pourtant aujourd'hui mis en question, comme l'a rappelé M. le ministre, par la directive européenne sur le temps de travail. Ce modèle d'engagement, envié dans le monde entier, qui irrigue toute notre société et que nous voulons conserver et transmettre aux générations futures, doit faire l'objet d'un combat mené aux côtés de plusieurs pays Plus que jamais, la balle est dans le camp du Gouvernement à ce sujet. Mais je suis rassuré par les propos du ministre de l'intérieur qui est déterminé à tirer parti de la prochaine présidence française du Conseil de l'Union européenne pour assurer des conditions de travail à la hauteur des sacrifices consentis par nos sapeurs-pompiers et pour consolider définitivement ce modèle de volontariat qui est véritablement la pierre angulaire de notre système de secours. secours. Ce rappel essentiel étant fait, si l'on en revient aux dispositions du texte, le Sénat a approuvé de nombreuses avancées de cette proposition de loi et a également participé à l'amélioration de son contenu au bénéfice des sapeurs-pompiers, acteurs locaux en lien permanent avec nos territoires. Je ne reviendrai pas sur les principales contributions de notre assemblée, qui ont été largement rappelées par notre rapporteure. Mais je tiens ici à saluer l'accord obtenu en commission mixte paritaire, qui reflète une volonté partagée par les deux chambres d'offrir aux acteurs de la sécurité civile les outils nécessaires, alors même que le champ de leurs missions tend à s'élargir et à devenir de plus en plus éprouvant. Sur ce sujet, nous avons pu transcender les clivages politiques. Qui pourrait penser que l'on perd ses convictions parce que l'on a le courage et la force de faire un bout de chemin ensemble ? Je suis très heureux que nous soyons parvenus à cette cohésion autour de notre modèle de sécurité civile. Tant de sujets ne devraient pas être abordés à travers le conflit traditionnel entre l'opposition et la majorité ! Je voudrais saluer ici la qualité du travail de nos rapporteurs, Françoise Dumont, Loïc Hervé et Patrick Kanner, qui ont oeuvré pour l'aboutissement du texte. Compte tenu des avancées offertes par cette proposition de loi qui consacre la modernisation de notre modèle de sécurité civile, notre groupe votera en faveur de ce texte, démontrant par là son attachement à une société de l'engagement propice à une véritable cohésion sociale.

nous devons beaucoup à ces héros du quotidien qui, souvent au péril de leur vie, viennent en aide à la population, combattent les incendies et tous les épisodes extrêmes de plus en plus nombreux et causés par le dérèglement climatique. L'accroissement majeur du nombre d'interventions durant ces dix dernières années n'est pas seulement dû à la crise sanitaire que nous vivons.

Dans cette optique, cette expérimentation nous apparaît cohérente et ses modalités plutôt rassurantes. Dans mon territoire d'ailleurs, une telle coordination existe déjà. Nous représentons les territoires et leur diversité, et nous serons attentifs aux conclusions de l'évaluation de ces expérimentations.

notamment au travers de la création du statut de pupille de la République pour les orphelins des pompiers décédés en service. Les pompiers et l'organisation des services d'incendie et de secours sont un maillon essentiel de notre République, une sorte de bras pacifique de la fraternité inscrite à notre devise républicaine. cette fraternité et cette solidarité, l'État doit leur octroyer les moyens leur permettant de préserver leur spécificité et d'exercer au mieux leurs missions. Aussi, malgré quelques réserves et quelques regrets, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires votera ce texte. La

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le 5 octobre dernier, un article de presse intitulé « Incendies : le drôle de statut des pompiers envoyés en renfort » revenait sur la situation révélée après les feux de forêt qui ont récemment eu lieu dans le Var. eu lieu dans le Var. Des centaines de pompiers professionnels, pour se relayer afin de lutter contre le feu, ont dû poser des congés et passer sous le statut de pompier

La présente proposition de loi ne donne pas de solution à ces problèmes de fond. Nous en avons supprimé l'article 22 A, qui n'avait pas d'impact sur la réglementation européenne fixant à 48 heures le temps de travail hebdomadaire maximum, et que nous ne pourrons pas continuer à contourner indéfiniment. Nous défendons avec force notre modèle de sécurité civile fondé sur le volontariat et l'engagement citoyen. Mais pour le préserver, il faut nécessairement mieux encadrer le statut de pompier volontaire, ce qui permettra également de le rendre plus attractif. La présente loi y contribue en partie, grâce à des revalorisations et à une plus grande reconnaissance, mais sans affronter le problème majeur. Cela implique également de renforcer les effectifs de pompiers professionnels, afin que les volontaires ne soient pas une simple main-d'oeuvre surutilisée, car financièrement plus rentable. Les remontées des SDIS sur ces pratiques sont faibles, alors qu'une plus grande transparence permettrait de mener un vrai travail à ce sujet. L'organisation d'assises nationales de la sécurité civile irait dans ce sens, surtout au regard des dernières mobilisations importantes des pompiers, qui dénoncent leurs conditions de travail et le manque de personnel. Les services d'incendie et de secours doivent faire face à des dépenses contraintes, à des interventions en augmentation, à une fragilisation des recrutements de volontaires alors que ces derniers représentent 79 % des pompiers, et à un financement par les départements qui connaissent des situations financières instables. Les défauts de moyens dans les services publics, comme dans les hôpitaux d'ailleurs, amènent les pompiers à aller au-delà de leurs missions et à combler ce recul de l'État, alors qu'ils sont eux-mêmes en sous-effectif chronique. Où sont les dispositions relatives aux effectifs et aux moyens financiers ? Je vous l'avais rappelé, le nombre de centres d'incendie et de secours chute, tout comme les dotations d'investissement. Nous voterons le texte élaboré

Le président Macron a annoncé le 16 octobre dernier que l'indemnisation des SDIS serait revalorisée et passerait de 124 euros à « au moins 200 euros » par carence. Nous espérons que cette promesse sera tenue, car une telle revalorisation est très attendue et apaisera les conflits entre SDIS et SAMU. Les débats demeurant autour des plateformes uniques montrent bien que la délimitation des compétences entre les différents acteurs de l'urgence demeure complexe, mais nous espérons que l'expérimentation permettra de dessiner des solutions, et nous sommes satisfaits que notre amendement visant à intégrer l'activité des plateformes déjà existantes à l'expérimentation ait été conservé dans le texte. Ces retours d'expérience sont précieux. Mais cette loi ne résoudra pas la situation de tension des services d'incendie et de secours. L'État doit être le garant de l'égalité des secours pour tous les citoyens, sur tout le territoire. Aujourd'hui, il faut de nouveaux moyens pour assurer cette proximité, mais également pour pour mieux protéger nos pompiers, qui sont de plus en plus victimes d'agressions. Les politiques d'austérité ou de surveillance appliquées depuis plusieurs gouvernements n'y répondent pas, pas plus que les mesures d'affichage comme la revalorisation de la prime de feu, en réalité financée par les départements. Cette proposition de loi a été votée à l'unanimité dans les deux chambres du Parlement. Elle nous réunit sur un sujet qui concerne la sécurité de toutes et de tous. Notre groupe votera cette loi, mais nous estimons qu'elle

réciproques - le Président de la République ne s'est pas trompé en les évoquant dans son discours lors du congrès des pompiers à Marseille, le 16 octobre dernier.

SAMU, pompiers, ambulanciers, téléalarme du département, Croix Rouge - et pourquoi pas, demain, monsieur le ministre, policiers et gendarmes ? -, tous ensemble pour servir nos concitoyens qui se trouvent dans une situation de détresse.

Cette vigilance pour les territoires se retrouve aussi dans la nécessité que les communes et les intercommunalités trouvent toute leur place dans la prévention des risques auxquels les populations sont exposées. La proposition de loi vient renforcer ces obligations.

on constate hélas que les violences contre les sapeurs-pompiers restent à un niveau élevé dans notre pays. Mes chers collègues, malgré les conditions difficiles d'examen de ce texte

Le cas est rare pour une loi qui compte 67 articles. Elle a été adoptée le 27 mai dernier à l'Assemblée nationale, alors que l'agenda parlementaire est contraint. Il faut saluer la performance et l'esprit de concorde.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous actons la suppression de l'article 22 A relatif à la réaffirmation du statut des sapeurs-pompiers volontaires, qui n'avait pas de portée normative, mais marquait un engagement commun de notre République. Vous avez, je crois, entendu notre souhait de voir résolus les problèmes liés à la directive du 4 novembre 2003 sur l'aménagement du temps de travail et à l'arrêt du 21 février 2018.

Nous prenons acte du fait que les dispositions relatives à l'anonymisation des plaintes déposées par des pompiers ne soient pas retenues dans le texte. Cela n'enlève rien à la qualité de la proposition de loi relative au renforcement de la sécurité des sapeurs-pompiers déposée par Patrick Kanner, adoptée ici le 6 mars 2019 à l'unanimité. Le travail sera poursuivi. J'en viens à un apport majeur de cette proposition de loi, qui changera tant la vie quotidienne de nos concitoyens que l'organisation territoriale du secours : la mise en place d'une plateforme commune, et son corollaire, la définition des carences ambulancières. Je me réjouis que la proposition de loi finale intègre les carences ambulancières constatées, comme le proposait le Sénat. Cette définition permet de consacrer l'étroit travail de concertation entre les SDIS et le SAMU, tout en prévoyant des dispositifs de secours.

Je partage pleinement l'analyse des sénateurs qui ont plaidé en commission mixte paritaire pour que les expérimentations ne soient pas établies au niveau régional, mais bien en intégrant directement l'échelon départemental. Il y va de l'efficacité même de l'expérimentation.

je souhaite que nous puissions ouvrir la question d'une part de péréquation dans les budgets des SDIS, afin de tenir compte des différenciations territoriales et des exigences de l'aménagement du territoire, cher à notre assemblée. Le groupe du RDSE sera favorable à cette proposition de loi.

le 127 congrès des sapeurs-pompiers qui s'est achevé il y a dix jours a montré quelles sont les attentes en matière de consolidation de notre modèle français de sécurité civile.

La sécurité civile appelle clairement un consensus politique. Par-delà la diversité de notre assemblée, nous y sommes parvenus, et je salue le texte qui nous est présenté aujourd'hui. L'engagement des sapeurs-pompiers est essentiel pour notre sécurité intérieure. Ce texte comporte des avancées notoires, qui vont dans le sens d'une reconnaissance, d'une adaptation et d'une pérennisation de l'engagement. Reconnaître l'engagement de nos sapeurs-pompiers, c'est d'abord reconnaître le service rendu par eux à notre République,

je suis heureux d'être aujourd'hui parmi vous pour débattre du projet de loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante, qui me tient particulièrement à coeur.

C'est un message que nous voulons collectivement envoyer à ces acteurs de l'économie de proximité et du quotidien. Le projet de loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante répond à un besoin impérieux de protection, de simplification et d'accompagnement des indépendants. Si le Gouvernement a pris depuis le début du quinquennat plusieurs mesures importantes en faveur des indépendants - je pense plus particulièrement au soutien à la création d'entreprise, à la réforme du régime social des indépendants, ainsi qu'à la création de l'allocation des travailleurs indépendants (ATI) il n'y a pas eu de projet global répondant à l'ensemble de leurs préoccupations. Ce projet de loi me tient aussi à coeur, parce que, depuis près de quarante ans, la défense des intérêts des indépendants m'anime au quotidien, pour des raisons d'équité, mais aussi et surtout pour des raisons de valeurs. Ces 3 millions d'indépendants, artisans, commerçants, professionnels libéraux notamment, qui ne comptent pas leurs heures et travaillent dur, illustrent des valeurs qui fondent notre pacte social : le mérite, le travail, la prise de risque et la volonté de transmettre.

malgré son ampleur et son caractère inédit, la crise que nous avons traversée au cours des dix-huit derniers mois n'a pas affecté ce dynamisme entrepreneurial. en 2020, le nombre total de créations d'entreprises a atteint un nouveau record, avec plus de 840 000 créations, soit 4 % de plus qu'en 2019, et cette tendance se confirme en 2021. Ce dynamisme entrepreneurial est important, car il reflète à la fois le niveau de confiance dans l'avenir et la dynamique créative du pays. Entreprendre, c'est une aventure formidable, mais la crise actuelle a souligné les risques qui pèsent sur les entrepreneurs et les difficultés que ceux-ci peuvent rencontrer tout au long de leur parcours. Nous ne pouvons plus nous satisfaire collectivement de cette situation. À la demande du Président de la République, nous avons préparé, durant une année, un plan qui, je le pense, répond aux attentes des indépendants. Ce plan, qui comprend une vingtaine de mesures, répond à un triple objectif protéger les indépendants face aux accidents de la vie ; mieux accompagner ces professionnels, de la création de l'entreprise à sa transmission ; simplifier les démarches. Le projet de loi qui fait l'objet des débats d'aujourd'hui est l'un des piliers de ce plan Indépendants,

Le projet de loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante que je vous soumets aujourd'hui permet tout d'abord la création d'un statut unique, protecteur du patrimoine personnel, pour l'exercice en nom propre d'une activité professionnelle. Les trois quarts des créateurs d'entreprises optent aujourd'hui pour le statut de l'entrepreneur individuel. De plus en plus jeunes- 41 % ont moins de 30 ans -et insuffisamment accompagnés, ces entrepreneurs individuels se rendent compte, souvent trop tard, que leur patrimoine personnel n'est pas protégé. août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a rendu la résidence principale insaisissable pour la liquidation des dettes professionnelles, il convient d'aller plus loin et d'étendre cette insaisissabilité à l'ensemble du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel. à cette protection, il sera mis fin au risque pesant sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel lorsque les difficultés professionnelles surviennent.

notamment à propos du transfert universel du patrimoine professionnel. Je suis persuadé que nous pourrons encore améliorer plusieurs dispositions du projet de loi en poursuivant nos échanges durant la navette parlementaire. Le Gouvernement ne soumettra donc pas, à ce stade, de nouvelle rédaction de l'article 1 du projet de loi.

Il s'agit d'une simplification majeure pour les créateurs d'entreprise, qui n'auront plus à choisir entre deux statuts pour l'exercice d'une activité en nom propre. En effet, le régime de l'EIRL, certainement trop complexe, n'a pas trouvé son public et son maintien ne sera plus justifié, car ses principaux avantages seront repris dans le nouveau statut. Enfin, la vie d'une entreprise implique parfois qu'un entrepreneur ait besoin de transmettre l'intégralité de son patrimoine à une autre structure. C'est le cas lorsqu'il a un projet de croissance et souhaite passer d'une entreprise individuelle à une société ; c'est également le cas lorsqu'il souhaite transmettre son entreprise à un tiers. Aujourd'hui, cette transmission est complexe, ce qui est parfois dissuasif. Les dispositions de ce projet de loi permettront aux indépendants de bénéficier d'un dispositif efficace du droit des affaires, donnant à ces professionnels la possibilité de transmettre la totalité de leur patrimoine professionnel en une seule opération, simple à réaliser.

l'allocation des travailleurs indépendants -, mais ce dispositif n'a été que très peu utilisé ; seules 1 000 allocations ont été accordées depuis la mise en place du dispositif. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de ce résultat. C'est pourquoi, dans le cadre du projet de loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante, nous proposons d'aller plus loin. Madame le rapporteur pour avis Puissat, je suis d'accord avec vous, la période de crise que nous traversons explique en partie ce faible recours au dispositif de l'ATI, les mesures d'urgence mises en place ayant permis aux indépendants de faire face aux difficultés économiques. ces mesures n'expliquent pas, à elles seules, ce résultat. Les conditions actuelles pour bénéficier du dispositif d'ATI sont très, voire trop, contraignantes et contribuent également à expliquer cette mesure où la plupart des indépendants cessent leur activité sans passer par une liquidation judiciaire ou par un redressement judiciaire, ils étaient exclus du dispositif. C'est pourquoi nous proposons que tout indépendant cessant son activité non viable puisse accéder, une fois tous les cinq ans, au dispositif de l'ATI. Un décret complétera la réforme de cette allocation, avec l'assouplissement du critère de revenu de 10 000 euros, qui ne sera désormais exigé que sur la meilleure des deux années. C'est une mesure d'assouplissement majeur, une plus équitable, qui permettra aux indépendants de préparer leur projet de reconversion tout en ayant un revenu de remplacement de 800 euros pendant six mois. Par ailleurs, la commission a adopté un amendement,

Je m'engage toutefois à ce qu'un rapport d'évaluation du dispositif soit remis au Parlement en 2024. En effet, je ne peux qu'adhérer à cette méthode de conduite des politiques publiques, qui s'appuie sur une évaluation régulière des dispositifs afin d'ajuster ces derniers aux besoins réels des entrepreneurs.

égard aux mutations majeures de notre économie, les dirigeants de PME ont besoin d'acquérir et de développer des compétences, afin de faire face, justement, à un environnement évoluant sans cesse. Or les indépendants ont encore très peu accès à la formation ; seuls 16 % d'entre eux ont bénéficié d'une action de formation financée par un fonds d'assurance formation en 2019.

projet de loi engage cette démarche, en procédant à la fusion des fonds d'assurance formation des artisans à partir du 1 janvier 2023. Avec cette réforme, les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale n'auront affaire qu'à un seul organisme chargé de la gestion de la contribution à la formation. Enfin, nous allons, dans le cadre de ce projet de loi, simplifier l'environnement juridique des indépendants grâce à l'adaptation de la procédure disciplinaire des experts-comptables, à la simplification du cadre juridique applicable aux professions libérales réglementées et à la rénovation du code de l'artisanat.

pour pouvoir concrétiser avant la fin du quinquennat l'ensemble des réformes comprises dans le plan Indépendants. Toutefois, la technicité des réformes proposées et la nécessité de poursuivre les consultations en cours nous obligent à passer par cette voie. La première ordonnance souhaitée par le Gouvernement tendait à adapter, à la suite de la réforme du statut de l'entrepreneur individuel, les dispositions relatives aux entreprises en difficulté et les dispositions relatives au surendettement des particuliers. La réforme proposée nécessite effectivement une mise en cohérence de plusieurs dispositions du code de commerce, du code rural et de la pêche maritime et du code de la consommation.

autorisant le Gouvernement à clarifier les règles communes applicables aux professions libérales réglementées, à simplifier et à adapter les différents régimes permettant aux professions libérales réglementées d'exercer sous forme de société et à faciliter le développement comme le financement des structures d'exercice des professions libérales, elle doit être, selon le Gouvernement, réintroduite dans le texte. La réforme que je vous propose aujourd'hui s'appuie notamment sur un rapport de l'inspection générale des finances, remis l'an dernier, elle a fait l'objet d'une première série de concertations avec les professionnels durant le premier semestre 2021. Toutefois, compte tenu de la technicité de la matière et de la diversité des professions libérales, j'ai souhaité poursuivre ces consultations afin d'ajuster les réformes en fonction des attentes et des besoins de chacune des professions. C'est pourquoi je propose de passer également par une ordonnance pour la mise en place de cette réforme. Je précise néanmoins qu'aucune modification, en matière de convergence des régimes ou de modulation des règles de détention du capital et des droits de vote, ne saurait être envisagée ni aboutir sans l'appui et l'accord formel des professions concernées. Enfin, la dernière ordonnance proposée vise à procéder à une nouvelle rédaction des dispositions du code de l'artisanat afin d'y intégrer les lois qui n'ont pas fait l'objet de codification. Il s'agit donc d'une mesure technique, menée à droit constant, qui n'apporte aucune modification de fond.

pour ce type de projet, afin de sécuriser la mise en place de cette réforme, plusieurs fois engagée, mais toujours reportée. En tout état de cause, je m'efforcerai, durant les débats, de vous apporter le plus de précisions possible sur le contexte de ces trois ordonnances. Monsieur le rapporteur Frassa, madame, monsieur les rapporteurs pour avis, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis persuadé que l'ensemble de ces mesures, complétées par des dispositions porteuses d'avancées significatives

d'échéances électorales importantes, un projet de loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante comportant diverses mesures d'inégale portée. Je me bornerai à évoquer celles qui relèvent de la compétence de la commission des lois, étant entendu que l'examen de plusieurs articles a été délégué à nos commissions des affaires économiques et des affaires sociales. La principale mesure de ce projet de loi consiste à soumettre l'ensemble des personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, en d'autres termes les « entrepreneurs individuels », à un nouveau régime juridique, qui déroge fortement, d'une part, au droit commun de la responsabilité civile et, d'autre part, au droit commun de la cession de biens et d'obligations. Vous le savez, l'un des principes fondamentaux de notre droit civil veut que toute personne qui contracte une dette vis-à-vis d'autrui réponde de cette dette sur l'ensemble de ses biens, présents et à venir. Comme le dit l'adage, « qui s'oblige oblige le sien ». Cette idée est au fondement de la notion de patrimoine, élaborée par Aubry et Rau au XIX siècle, dont la fonction première est d'asseoir la responsabilité de la personne vis-à-vis des tiers. Il en résulte un principe d'unicité du patrimoine : diviser celui-ci reviendrait en effet à priver chacun des créanciers d'une partie de son gage. Depuis fort longtemps, les pouvoirs publics ont apporté des tempéraments à ces principes, afin de protéger les entrepreneurs et les investisseurs contre les aléas de la vie économique. Ce fut d'abord la raison d'être des sociétés commerciales à responsabilité limitée, qui, depuis une loi du 11 juillet 1985, peuvent être constituées d'un seul associé. tous les entrepreneurs n'exercent pas sous forme sociétaire. Environ 3 millions de personnes exercent aujourd'hui, en France, une activité professionnelle indépendante en leur nom propre. Pour les protéger, le législateur a cherché à soustraire leurs biens les plus précieux aux poursuites de leurs créanciers professionnels. Ce fut d'abord le cas de leur résidence principale, puis éventuellement d'autres biens immobiliers à usage non professionnel, qui peuvent être rendus insaisissables. Une loi du 15 juin 2010, due à l'initiative du secrétaire d'État Hervé Novelli, est allée plus loin, en ouvrant une première brèche dans le principe d'unicité du patrimoine : c'est le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou EIRL. Ce régime permet à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante d'affecter à cette activité un patrimoine distinct de son patrimoine personnel. Ses créanciers professionnels n'exercent alors leur droit de gage général que sur son patrimoine affecté, ses créanciers personnels le faisant sur son patrimoine non affecté. Le bénéfice du régime de l'EIRL est soumis à un formalisme assez lourd, qui a pour objet de garantir la sécurité juridique de l'entrepreneur et des tiers. C'est sans doute ce qui explique, au moins en partie, que ce régime n'ait pas eu le succès escompté, puisque l'on ne compte aujourd'hui qu'un peu moins de 100 000 EIRL. L'article 1 du présent projet de loi va beaucoup plus loin, en prévoyant que, dorénavant, toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante serait titulaire de plein droit de deux patrimoines, l'un professionnel, l'autre personnel. La délimitation des deux patrimoines résulterait non plus d'une déclaration d'affectation assortie d'un inventaire, mais d'un simple critère légal : l'utilité des biens, droits ou obligations pour l'activité professionnelle indépendante de la personne concernée. En principe, le gage général des créanciers professionnels et personnels serait limité au patrimoine correspondant, mais ce principe connaîtrait des exceptions. Le projet de loi prévoit ainsi que l'entrepreneur individuel pourra renoncer au bénéfice de la séparation des patrimoines en faveur d'un créancier et à l'occasion d'un engagement déterminé : il répondrait alors de sa dette sur l'ensemble de ses biens. Le texte du Gouvernement prévoyait aussi de larges dérogations au profit de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale, que nous avons réduites à de plus justes proportions. Par ailleurs, le patrimoine professionnel pourrait être transmis entre vifs, à un tiers, en tant qu'universalité. Il s'agit notamment de faciliter la transformation de l'entreprise individuelle en société, mais cela exigera aussi une modification des règles fiscales, aujourd'hui très défavorables à cette opération. Il s'agit d'une réforme indéniablement audacieuse et nous pouvons, selon moi, souscrire à ses objectifs. Beaucoup d'entrepreneurs individuels expriment le besoin d'être mieux protégés contre les conséquences d'un échec. Renforcer leur protection, c'est aussi stimuler l'initiative économique. Néanmoins, il nous faut être prudents si nous ne voulons pas réduire à néant le crédit des entrepreneurs individuels. Il ne faut d'ailleurs pas s'exagérer les effets réels de cette réforme sur la protection des biens des entrepreneurs individuels, car les créanciers les plus importants, notamment les banques, exigeront désormais systématiquement des sûretés spéciales sur certains biens, voire une renonciation pure et simple au bénéfice de la séparation des patrimoines Par ailleurs, le texte du Gouvernement présentait des lacunes et des fragilités juridiques, dont les conséquences pouvaient être très fâcheuses, pour les entrepreneurs individuels eux-mêmes comme pour les tiers. La commission s'est attachée à les corriger. L'une de nos divergences avec le Gouvernement tient à la conception que nous nous faisons du domaine de la loi. Des pans entiers du nouveau statut de l'entrepreneur individuel, indispensables pour garantir la sécurité juridique de la réforme, sont renvoyés, dans le texte du Gouvernement, à un décret en Conseil d'État. C'est, pour nous, inacceptable. Le Conseil d'État a lui-même laissé entendre que le Gouvernement méconnaissait ainsi l'article 34 de la Constitution, qui réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux du droit de propriété et des obligations civiles et commerciales. Il ne s'agit pas pour nous de défendre notre pré carré de faire respecter cette garantie, liée, pour les citoyens, au fait que certaines règles touchant de près à l'exercice des droits et libertés ne peuvent être fixées que par la loi, c'est-à-dire, en principe, du moins, par les représentants élus de la Nation et après un débat public. Je ne voudrais pas que le Gouvernement, après avoir usé et abusé des ordonnances, recherche à présent un autre moyen de contourner le Parlement en vidant de sa substance le domaine de la loi Il se heurterait, en tout état de cause, au Conseil constitutionnel, qui censure invariablement l'incompétence négative du législateur. À l'article 4, la commission des lois a supprimé la demande d'habilitation, visant à tirer, par voie d'ordonnance, les conséquences du nouveau statut de l'entrepreneur individuel sur les procédures collectives et les procédures de surendettement des particuliers, d'y substituer des dispositions d'application directe. L'article 6 comportait une autre demande d'habilitation à légiférer par ordonnance, pour modifier les règles applicables à l'exercice en société des professions libérales réglementées. La commission des lois l'a supprimé, car le sujet est beaucoup trop sensible pour que le Parlement abandonne sa compétence. Nous devons en particulier veiller à préserver les règles visant à garantir l'indépendance des professionnels libéraux qui exercent au sein d'une société, qu'il s'agisse des règles de composition du capital ou des règles relatives à la répartition des droits de vote. Je passe plus rapidement sur l'article 8, qui prévoit que les dettes professionnelles sont prises en compte pour l'appréciation de la situation d'une personne qui demande l'ouverture d'une procédure de surendettement des particuliers.

réforme le régime disciplinaire des experts-comptables pour tenir compte, notamment, de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui impose la séparation des fonctions de poursuite et de jugement et prohibe la révocation automatique du sursis, en cas de nouvelle condamnation.

et s'est également vu déléguer au fond l'examen de deux articles, l'article 7, qui traite du code de l'artisanat, et l'article 12, relatif au dialogue social au sein des chambres de commerce et d'industrie Alors que les grandes entreprises et les PME ont bénéficié d'une succession de plans ces dernières années, les travailleurs indépendants, eux, ont souvent été laissés de côté. Le dernier texte les concernant au premier chef remonte à 1994. Aucun plan exhaustif et structurant n'a, depuis lors, vu le jour.

bien qu'ils ne soient pas les seuls touchés, il ne peut être nié que ces professionnels font face à une succession de crises importantes depuis plusieurs années. Or ces entrepreneurs sont dans une situation fragile : la crise a diminué leur revenu d'activité et a conduit une partie d'entre eux face à un mur d'endettement. Les lendemains de crise risquent donc d'être particulièrement difficiles ... En outre, les travailleurs ayant opté pour le statut d'entrepreneur individuel sont responsables sur l'intégralité de leur patrimoine.

En dépit de ces motifs de satisfaction, plusieurs incertitudes ne sont pas levées par le projet de loi. Par exemple, il est à peu près certain que les créanciers, au premier rang desquels figurent les banques, ne se satisferont pas de la situation et qu'elles exigeront de l'entrepreneur qu'il renonce expressément à la protection de son patrimoine personnel. Dans les faits, donc, l'entrepreneur n'aura finalement que peu de choix, puisqu'il risquera de perdre son financement. De même, nous craignons que la simplicité recherchée soit plus que compensée par les nombreuses demandes de garanties qui émaneront des créanciers. J'en viens maintenant aux deux articles délégués au fond à notre commission. L'article 7 est une habilitation à légiférer par ordonnance tendant à clarifier, à droit constant, la rédaction et le plan du code de l'artisanat. Nous avons choisi, malgré nos réserves à l'égard des ordonnances, de ne pas nous opposer à celle-ci

Cela signifie donc que le personnel de droit privé, bien qu'il représente maintenant un tiers des effectifs de ces organismes, n'est pas représenté, alors même que la négociation porte sur une convention qui le concerne au premier chef. Cet article inverse donc la situation, en prévoyant des élections six mois après la publication de ce texte et en fixant une période d'un an et demi de négociations pour parvenir à la signature de la convention. Si celle-ci n'est toujours pas adoptée, c'est la convention collective des métiers du conseil et de l'accompagnement aux entreprises qui s'appliquera. Il nous semble que ces dispositions sont de nature à sortir de l'impasse. La commission a toutefois précisé que, en cas d'élection partielle dans l'une des 18 CCI, le résultat de celle-ci ne pourra être invoqué pour provoquer de nouvelles élections générales dans les 17 autres, la représentativité syndicale étant calculée à partir de la dernière élection générale et pour toute la durée du cycle électoral, c'est-à-dire quatre

L'article 9 porte sur l'allocation des travailleurs indépendants, instituée par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, afin de couvrir les travailleurs non salariés contre le risque de perte d'emploi. Le dispositif est applicable depuis le 1 novembre 2019. Cette prestation, d'un montant forfaitaire de 800 euros par mois et intégralement financée par l'assurance chômage, mais non contributive, est versée pendant une période maximale et non renouvelable

Les indépendants contribuent donc à hauteur de 14 % au budget de cet organisme. Cela doit nous inviter à nous interroger plus largement sur la gouvernance de l'assurance chômage. L'ouverture de ce nouveau droit a toutefois été très prudente et les conditions pour en bénéficier sont restrictives.

Nous sommes donc loin de l'assurance chômage universelle annoncée ! Dans ce contexte, l'article 9 vise à ouvrir une nouvelle voie d'accès à l'ATI, en ajoutant une condition alternative à la cessation d'activité définitive et involontaire sanctionnée par une procédure de liquidation judiciaire ou un plan de redressement judiciaire auraient ainsi droit à l'ATI les travailleurs dont l'entreprise a fait l'objet d'une déclaration de cessation totale et définitive d'activité, lorsque cette activité n'est pas viable économiquement. Cet article tend également, afin de prévenir l'aléa moral que pourrait engendrer cette ouverture, à mettre en place un délai de carence de cinq ans entre deux demandes d'ATI. L'attente croissante de protection sociale de la part des travailleurs indépendants, en lien avec l'avènement des microentrepreneurs, plaide pour ouvrir les conditions d'accès au dispositif. On peut toutefois s'interroger, à la suite de nos collègues rapporteurs, sur la temporalité de la réforme proposée, qui intervient après moins de deux ans de fonctionnement de la prestation, dont quatre mois seulement ont été significatifs en raison de la crise sanitaire. Cette réforme précoce, en l'absence de véritable bilan, selon la commission des affaires sociales, l'introduction d'une véritable « clause de revoyure », après concertation avec les partenaires sociaux et les représentants des travailleurs indépendants. faut marcher sur ses deux jambes, la commission a également proposé que les travailleurs indépendants soient informés de la possibilité de souscrire un contrat d'assurance complémentaire contre la perte d'emploi subie ainsi que du dispositif « Madelin » de déduction fiscale. L'article 10 est relatif aux circuits de financement de la formation professionnelle des travailleurs indépendants, et notamment des artisans. Il vise à remédier à une anomalie historique. En effet, les chefs d'entreprise artisanale sont les seuls travailleurs non salariés qui dépendent de deux guichets pour le financement de leur formation professionnelle d'une part, les conseils de la formation (CDF), au sein des chambres régionales de métiers et de l'artisanat (CRMA) ; d'autre part, le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale (Fafcea). Le système est peu efficient et l'existence de deux guichets est source de complexité pour les professionnels concernés. Par ailleurs, les ressources des fonds de la formation professionnelle des artisans ont radicalement diminué à la suite du transfert, en 2018, de la collecte de la contribution En particulier, les nombreuses erreurs de fléchage constatées depuis cette réforme ne semblent pas encore résolues. L'article 10 prévoit d'unifier le financement de la formation professionnelle des artisans en affectant les sommes collectées à un unique fonds d'assurance formation de droit commun. harmonise plus largement les circuits de financement de la formation des travailleurs indépendants en confiant à France compétences la répartition des sommes collectées entre les différents affectataires. Cette évolution répond à une attente de simplification des professionnels concernés. Elle suscite néanmoins certaines inquiétudes. Sans remettre en cause la plus grande souplesse que devrait permettre l'unification des fonds, la commission des affaires sociales a proposé d'associer le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat à la gouvernance du futur fonds unique. Afin de prévenir le risque de ruptures de financement semblables à celles que les fonds ont subies en 2019 du fait d'une réforme insuffisamment préparée, la commission a également adopté, à l'article 14, un amendement visant à reporter au 1 janvier 2023 l'ensemble de la réforme. est, mes chers collègues, l'avis de la commission des affaires sociales sur ce texte. Il resterait beaucoup à faire, notamment en matière d'équité du prélèvement et de la protection sociale entre salariés et indépendants. Toutefois, ce texte a le mérite de mettre en lumière les problématiques spécifiques d'une catégorie souvent oubliée. Il est donc important, comme l'a souligné M. le rapporteur, de le voter. La parole est à M.

en 1979, Michel Foucault prononçait au Collège de France un cours intitulé. Il y retraçait l'histoire du libéralisme, depuis l'émergence de l'économie politique au XVIII siècle jusqu'à l'avènement de l'entrepreneur en tant qu'archétype de l'individu moderne. Selon Foucault, cet individu moderne est en effet devenu l'entrepreneur de lui-même. Par le travail qu'il effectue et par les risques qu'il prend, il développe son capital personnel. Dans nos sociétés libérales, la quête de l'autonomie est donc le résultat d'un processus culturel et politique au long cours. C'est ainsi que la figure de l'entrepreneur s'est imposée comme un modèle d'accomplissement, qui dépasse largement le cadre de l'activité professionnelle. Être entrepreneur, ce n'est pas avoir un statut, c'est se rendre maître de sa vie. Et pourtant, les indépendants, qui n'ont pas attendu le cours de Foucault pour mettre la main à la pâte, aimeraient bien que leur statut soit mieux reconnu. Il faut les comprendre : de même que nos politiques économiques sont toujours taillées sur mesure pour les grandes entreprises, nos politiques sociales, elles, sont taillées sur mesure pour les salariés. Autrement dit, les indépendants, qu'ils soient artisans, libéraux, commerçants ou patrons de PME, n'entrent jamais dans les bonnes cases, car les cases ne sont pas toujours faites pour eux. C'est tout le paradoxe de la France : d'une part, on y fait l'éloge des citoyens qui deviennent les entrepreneurs d'eux-mêmes ; d'autre part, on décourage sans cesse les indépendants, en dressant sur leur parcours mille et un obstacles administratifs. C'est précisément ce paradoxe qui se trouve à l'origine du projet de loi que nous examinons aujourd'hui. Ce texte vise à la fois à simplifier et à sécuriser le parcours des indépendants, du début jusqu'à la fin de leur activité, en envisageant aussi les cas où tout ne se passe pas comme prévu, voire se passe carrément mal. L'échec demeure en France le grand tabou, si bien qu'il est souvent peu et mal traité par nos lois. Or si l'individu devient, dans tous les aspects de sa vie, l'entrepreneur de lui-même, tous les aspects de sa vie ne doivent pas se réduire à son activité professionnelle et, éventuellement, à son échec. C'est pourquoi l'article 1 du projet de loi, qui redéfinit le statut de l'entrepreneur individuel et distingue le patrimoine professionnel du patrimoine personnel, me paraît tout à fait essentiel. L'entrepreneur qui investit son capital prend déjà son risque ; il n'est pas juste qu'il doive en outre hypothéquer sa maison et ses économies pour tenter sa chance. De même, l'article 9, qui vise à élargir les critères de l'allocation des travailleurs indépendants, la trop peu fameuse ATI, contribue à adapter notre modèle social aux caractéristiques de l'activité indépendante. Cette allocation n'a pas encore trouvé son public : non pas que les indépendants n'en aient pas éprouvé le besoin, surtout en ces temps difficiles,

l'entrepreneur qui a connu l'échec doit pouvoir compter sur une aide d'urgence, sans attendre une procédure de liquidation judiciaire. Toujours en matière de simplification, la mise en extinction du statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée sera d'une aide précieuse pour tous les futurs entrepreneurs. Force est de constater que les avantages de l'EIRL n'ont pas eu raison de sa complexité. Ce statut demeurait trop peu attractif et nuisait, de manière générale, à la lisibilité des différentes options qui s'offrent aux créateurs d'entreprises. Le transfert des avantages de l'EIRL vers un statut unique simplifiera donc la vie des Français qui font le choix de se mettre à leur compte. Ces mesures, d'apparence technique, ont le grand mérite, au pays des complexités administratives et fiscales, de simplifier la vie des indépendants. Et vous le savez mieux que quiconque, monsieur le ministre, ils demandent non pas qu'on fasse plus pour eux, mais simplement qu'on les laisse travailler en paix. C'est pourquoi je me réjouis que le Gouvernement ait inscrit ce texte à l'agenda parlementaire. Je suis sûr qu'il contribuera, de manière très concrète, à simplifier la vie des entrepreneurs et à sécuriser leur activité tout au long de leur parcours. La relance ne se fera pas sans le concours de nos artisans, de nos commerçants, de nos autoentrepreneurs, de nos professions libérales, bref, de tous les indépendants qui font vivre en France les valeurs de travail et d'autonomie. Ils ont tenu bon pendant la crise ; ils sont aujourd'hui aux avant-postes de la reprise. Et s'ils sont aujourd'hui essentiels à notre économie, ils le seront encore plus demain. Les jeunes générations ne rêvent plus d'une carrière faite d'un emploi salarié au sein d'une même entreprise. Elles aspirent à la multi-activité, sans avoir à choisir de façon définitive entre salariat ou entrepreneuriat. Nous ferons donc oeuvre utile pour les futures générations en adaptant notre modèle social à ces nouvelles aspirations et à ces nouvelles formes de travail. Il s'agit en effet de permettre à chaque citoyen de devenir l'entrepreneur de lui-même.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui un projet de loi important, puisqu'il tend à répondre au développement inédit de nouvelles formes d'organisation et de modalités du travail. Sans même évoquer les effets de la crise sanitaire, le marché du travail connaît des mutations profondes. Surtout, les aspirations d'un nombre toujours plus grand de nos concitoyens évoluent nettement, singulièrement celles des jeunes générations pour lesquelles le salariat, dans sa conception traditionnelle, n'est plus un choix automatique. Dès lors, la création d'un nouveau statut unique de l'entrepreneur individuel a des implications importantes, et ce d'autant plus qu'elle devrait concerner près de 2,8 millions de travailleurs, hors secteur agricole.

Nous saluons la nouvelle rédaction de l'article 1, qui permet d'éviter un certain nombre de conséquences pouvant s'avérer préjudiciables tant pour les entrepreneurs individuels que pour les tiers. Tel est le cas, notamment, du critère choisi pour assurer la démarcation entre les deux patrimoines de l'entrepreneur individuel : l'instauration de règles de preuve nous semble ici plus à même d'apporter de la sécurité à l'entrepreneur individuel comme à ses créanciers. Dans le même sens, la proposition du rapporteur d'encadrer davantage les exceptions à la séparation des patrimoines, dont bénéficieraient à la fois les services fiscaux et ceux de la sécurité sociale, est particulièrement pertinente si l'on souhaite que la réforme se traduise par des résultats concrets pour les entrepreneurs individuels. Naturellement, nous souscrivons aux différentes initiatives du rapporteur visant à supprimer les habilitations du Gouvernement à légiférer par ordonnance, notamment celle qui ambitionnait de réformer le droit applicable à l'exercice en société des professions libérales réglementées. Cette question est bien trop sensible pour que le Parlement ne puisse, en tant que législateur, y apporter pleinement son concours. Enfin, il nous semble nécessaire de permettre aux acteurs économiques concernés, en particulier les banques, de s'adapter à cette nouvelle réglementation. L'entrée L'entrée en vigueur du nouveau statut de l'entrepreneur individuel gagnera pleinement à être différée de trois mois. Il en va de même de la mise en extinction du régime de l'EIRL. Pour conclure, je remercie notre rapporteur de la commission des lois, ainsi que nos collègues Frédérique Puissat et Serge Babary, de la qualité de leur travail. Je ne doute pas que les sénateurs du groupe Les Républicains voteront ce projet de loi, tel qu'il sera amendé par notre assemblée. La parole est à Mme Mélanie

Mme Mélanie Vogel. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi s'inscrit dans le plan en faveur des travailleurs indépendants, annoncé par le Président de la République à la fin du mois de septembre dernier, et comporte différentes mesures de portée inégale. Les indépendants recouvrent des situations très variées et regroupent un grand nombre de métiers du quotidien, qui vont du commerçant et de l'artisan aux professions libérales, en passant par les travailleurs des plateformes. Les obstacles qu'ils doivent surmonter sont multiples. Nombre d'entre eux ont été durement touchés par la crise sanitaire et sociale,

La principale mesure du texte consiste en la création d'un nouveau statut de l'entrepreneur individuel, aux termes duquel le patrimoine personnel devient par défaut insaisissable par les créanciers. Seuls les éléments nécessaires à l'activité professionnelle pourront être saisis en cas de défaillance. Compte tenu de Compte tenu de la situation économique, de plus en plus d'indépendants font face au risque majeur de voir leurs dettes professionnelles recouvrées en partie sur leur patrimoine personnel. Cette disposition est plutôt bienvenue pour mieux les protéger contre les conséquences d'un échec. Cependant, nous pouvons assez facilement penser que les créanciers demanderont à l'entrepreneur de renoncer expressément à la protection de son patrimoine personnel ou, comme l'a souligné M. le rapporteur pour avis, demanderont des sûretés conventionnelles.

nous proposerons un amendement visant à conditionner la création d'une entreprise individuelle à la réalisation d'une étude préalable de marché, soumise aux chambres de commerce et d'industrie, qui rendront un avis non contraignant sur l'opportunité et la solidité de chaque projet d'entreprise. Cela permettrait d'éviter de laisser entrer sur le marché des personnes en situation de grand risque. situation de grand risque. L'article 12 apparaît comme un cavalier eu égard à l'objet du texte : cet article prévoit en effet de modifier des dispositions transitoires, déjà fragiles, prévues dans la loi Pacte, en inversant l'ordre procédural actuel en matière d'élections syndicales et de négociation de la convention collective des personnels de droit privé au sein du réseau des CCI des CCI sans que le dialogue social ait pu être mené à terme. Définir l'entrée en vigueur d'une convention collective non aboutie sur de nombreux sujets majeurs, comme l'égalité femme-homme, le congé de paternité ou encore le forfait jour, est une curieuse conception du dialogue social. C'est pourquoi nous proposerons la suppression de cet article.

Nous regrettons que ce projet de loi ne réponde pas aux enjeux des nouvelles formes de travail. Il passe totalement sous silence la question de l'« ubérisation » et des difficultés que rencontrent les travailleurs indépendants des plateformes numériques, qui peuvent constituer une nouvelle forme d'exploitation. Votre ordonnance sur les modalités de représentation des travailleurs des plateformes ne va pas beaucoup plus loin. Emmanuel Macron avait axé sa campagne sur le travail, la liberté d'entreprendre et les protections sociales qui doivent accompagner les mutations du salariat qui sont en cours. Nous entendons les aspirations d'une partie de la population, notamment de la jeunesse, qui peut être séduite par ces nouvelles formes de travail non salarié : exercer son métier de manière autonome, choisir ses modalités d'organisation, son rythme de travail, ses horaires, ne pas être dans une situation de subordination, tout cela a beaucoup d'attraits. C'est aussi une prise de risque, qui doit être assumée et décidée en toute connaissance de cause. Mais, cinq ans après, si peu a été fait vous n'avez pas ouvert l'indemnisation du chômage à tout le monde, comme vous l'aviez promis, mais seulement aux démissionnaires ; vous n'avez pas construit la protection sociale des travailleurs des plateformes, mais seulement une allocation des travailleurs indépendants, perçue par moins de 1 000 personnes vous n'avez presque rien fait pour empêcher le détournement du statut d'autoentrepreneur en salariat déguisé ; vous n'avez pas non plus imaginé la participation de ces activités à l'effort de protection sociale. Plus largement, c'est la philosophie globale de ce projet qui nous amène à nous interroger. Ce texte illustre le renoncement croissant de la puissance publique à oeuvrer pour bâtir l'environnement macroéconomique favorable à la création de l'emploi et qui préfère se défausser sur les individus qui ont la charge de créer leur propre activité. Un tel renoncement devrait vous conduire à épouser les thèses de nombreux économistes et responsables politiques sur la nécessité de construire un revenu universel, pendant indispensable d'une telle responsabilité individuelle- mais il n'est en rien.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues,

Il s'agit d'alléger encore les formalités de création d'entreprise ce nouveau statut d'entrepreneur individuel et l'extension de l'allocation des travailleurs indépendants, cette prestation « mal née » qu'ils ne demandaient pas, pour reprendre les mots de la commission des affaires sociales. Ce texte concernera près de 3 millions de personnes- commerçants, artisans, professions libérales, professionnels du spectacle, entrepreneurs agricoles ... Encore une fois, monsieur le ministre, nous observons un décalage entre les besoins des entrepreneurs et les mesures proposées. S'il apparaît effectivement important de mieux protéger les travailleurs indépendants, la scission des patrimoines personnels et professionnels de l'entrepreneur nous interroge à plusieurs titres et nous laisse penser qu'il s'agit d'une mesure d'affichage. En effet, le formalisme, les procédures servent à protéger l'entrepreneur et les tiers. Il en est ainsi de la description, sous forme d'inventaire, de ce qu'est le patrimoine professionnel- inventaire qui sera d'ailleurs supprimé et remplacé par une définition légale aux contours assez flous. Comme cela a été souligné lors des débats en commission, la notion d'« utilité », qui servira de ligne à la séparation des deux patrimoines, risque d'être élargie au maximum par les créanciers. De plus,

la limite de ce texte : l'entrepreneur pourra renoncer à la scission de son patrimoine à la demande d'un créancier. Dans ce cadre, comment ignorer que les créanciers les plus importants exigeront de l'entrepreneur qu'il renonce expressément à la protection de son patrimoine personnel ou demanderont des sûretés conventionnelles ? Dans les faits, il n'aura guère le choix. En ce sens, ce projet de loi n'apporte pas de réponse claire aux problèmes réels des entrepreneurs individuels. Le texte ne contient aucune obligation à la charge des banques et ne mettra pas fin à leurs pratiques actuelles. Pour notre part, nous renouvelons ici notre proposition de créer une banque publique offrant des prêts à taux zéro pour accompagner

il est proposé de mettre en place un « délai de carence » entre deux demandes. Ainsi, une personne ne peut bénéficier de l'ATI pendant cinq ans à la suite d'une défaillance. Or on peut se demander s'il ne serait pas plus opportun d'aider un entrepreneur à sortir d'un statut qui ne lui convient pas

pas. C'est d'un accompagnement véritablement pédagogique que les aspirants entrepreneurs ont besoin. En ce sens, la suppression du stage de préparation à l'installation est pour nous une erreur, car il est important d'avoir une formation minimale à la gestion d'entreprise, notamment en matière de fiscalité et de régimes sociaux. Très bien ! Il est aussi essentiel de trouver des informations sur les entreprises récemment créées, sur les secteurs porteurs. Par exemple, le pourcentage des entreprises qui survivent au-delà de la première année ? De même, la question du financement et du rôle des banques n'est pas abordée, alors que l'échec des réformes de l'entrepreneuriat individuel s'explique aussi par la par la frilosité des banques à financer les entrepreneurs. Aucune charte ne pourra obliger les banques à jouer leur rôle de financement tout en acceptant la séparation des patrimoines. le texte oublie les travailleurs victimes de l'ubérisation, faux indépendants compte tenu des liens de subordination qui les unissent à leurs employeurs. Nous savons pourtant tous que le statut d'autoentrepreneur permet à certains de contourner les garanties du salariat et de faire l'économie des cotisations patronales. Enfin, rien sur la baisse de pouvoir d'achat des Français, qui emporte nécessairement des conséquences Comme le disait en 2010 mon amie Nicole Borvo à propos de la création de l'EIRL : « Le projet de loi qui nous est aujourd'hui soumis affiche une bonne intention : réformer le statut de l'entrepreneur individuel pour le protéger, lui et sa famille, contre les conséquences désastreuses d'une faillite ; il est loin, je le crains, de tenir ses promesses. » Je crois qu'elle n'avait pas tort. Aujourd'hui, sous le prétexte de libérer le travail et d'agir dans l'urgence, le Gouvernement est en train de créer un statut

Balzac décrit à merveille cette triste réalité humaine. L'esprit de ce texte se résume à ces deux mots : protéger et simplifier.

le besoin d'être mieux protégés. Il est essentiel que les conséquences d'un échec dans le lancement d'une activité entrepreneuriale ne remettent pas en cause l'équilibre financier de toute une famille, de toute une vie parfois. Nous espérons aussi que cela pourra stimuler l'activité économique et finir de convaincre ceux qui hésitent encore à se lancer, de peur des conséquences financières. La situation économique des entrepreneurs a été fragilisée ces temps derniers par plusieurs crises successives-

Grâce à cette disposition, le passage de l'exercice d'une activité en nom propre à une société sera fluidifié, ce qui permettra de faciliter la croissance et la transmission des entreprises. Tout ce qui va dans le sens de la simplification est une bonne chose. L'un des exemples ultimes en la matière étant la création du statut d'autoentrepreneur. Ces dispositions vont dans le bon sens. Toutefois, le groupe Union Centriste, à l'instar des trois commissions saisies de ce texte, constate encore plusieurs zones d'ombre qu'il nous faudra éclairer ensemble. Tout d'abord, il ne faut pas que cette nouvelle protection soit

Sur ce point, je rejoins notre collègue rapporteur Serge Babary : les banques ne se satisferont pas d'un droit de gage ne portant que sur le patrimoine

Pour répondre à cette inquiétude, notre groupe partage et soutient la proposition du rapporteur, qui appelle le Gouvernement et les banques à élaborer une charte d'engagement quant aux conditions de financement des entrepreneurs individuels. Cet engagement important permettra d'assurer la pérennité du projet de loi. Notre seconde inquiétude est liée à l'article 6 et, plus généralement, à la volonté du Gouvernement de légiférer par ordonnance. Le groupe Union Centriste rejoint

Notre groupe est très attentif au respect du Parlement, de ses élus comme du débat en son sein. Il nous revient de légiférer en tant que représentants du peuple et des collectivités. Je le dis souvent aux maires que je rencontre dans mon département, comme hier soir : le Sénat n'est pas le. Il est

enfin lancer une alerte sur l'article 10. Pour des raisons historiques, les chefs d'entreprise artisanale et les microentrepreneurs inscrits au répertoire des métiers sont les seuls travailleurs non salariés qui dépendent de deux guichets

pouvez-vous nous assurer que cette modification du circuit de financement de la formation de ces professionnels ne se traduira pas par des déperditions ? Les difficultés de fléchage rencontrées par les Urssaf ne sont pas résolues Par ailleurs, la situation financière de France compétences nous inspire des doutes quant à l'opportunité d'un transfert à cet opérateur de la répartition de nouveaux flux et fait craindre des dommages pour les acteurs concernés.

la situation des professionnels indépendants- cela a été dit -est très contrastée. Ils ou elles exercent leurs activités dans des secteurs économiques variés : agriculture, artisanat, commerce, professions libérales, mais aussi plateformes numériques, le statut de travailleur indépendant Le principal enjeu d'un tel projet de loi est de fixer des règles communes et intelligibles pour un état professionnel qui n'a pas de définition unique. Il existe plusieurs statuts d'entreprise individuelle, plusieurs régimes de protection sociale, plusieurs secteurs d'activité, etc. Du point de vue financier, entre le revenu moyen d'un indépendant, situé autour de 2 500 euros net mensuels, et celui d'un microentrepreneur, plus proche de 500 euros, il y a un monde ... Même chez les indépendants bénéficiant de revenus corrects, on peut rencontrer des L'ambition affichée est de répondre à une multiplicité de questions : simplification des statuts juridiques, amélioration de la protection sociale, sécurisation du patrimoine personnel, meilleure formation Le texte semble y pourvoir en partie, avec la réécriture des dispositions du livre V du code de commerce relatives au statut de l'entrepreneur individuel, mais aussi des mesures institutionnelles comme la fusion des fonds d'assurance des artisans, le renforcement des procédures disciplinaires applicables aux experts-comptables ou encore, quoique le lien paraisse moins évident, le mode de gestion des chambres de commerce et d'industrie. La commission des lois a effectué des modifications substantielles, en réécrivant complètement certains articles qui sont au coeur du dispositif et en supprimant ou restreignant le champ des trois habilitations prévues dans la version initiale. Elle a également inséré dans le texte de nouvelles dispositions

estimé que cette mesure, en l'état, n'avait pas sa place dans le présent projet de loi ; c'est pourquoi j'en proposerai la suppression. L'entrée en vigueur de la plupart des mesures a également été reportée. Mon groupe s'est penché de son côté, depuis plusieurs mois, sur cette question des indépendants et a saisi l'occasion de l'examen de ce projet de loi pour attirer l'attention sur certains sujets à mon sens relativement urgents, comme ceux des garanties personnelles exigibles en cas d'emprunt bancaire ou de la dématérialisation et de la simplification des procédures administratives. Aujourd'hui encore, les professionnels indépendants sont trop souvent confrontés à des difficultés lorsqu'ils souhaitent réaliser des projets d'investissement ; ils doivent apporter des garanties qui font peser une lourde hypothèque sur leurs biens personnels. Pour encourager l'esprit d'entreprise, il faut que les risques soient équitablement répartis. C'est pourquoi je regrette, à l'instar de mes collègues, un certain manque de visibilité et de lisibilité de ce projet de loi, qui contient des mesures essentiellement techniques et arrive en fin de législature, alors que la situation des indépendants fait l'objet de discussions et de propositions depuis plusieurs années-

Gardons aussi à l'esprit qu'il s'agit d'un ensemble de professions qui sont souvent éloignées, par construction, du monde administratif, et pour lesquelles l'idée de réglementation ne va pas nécessairement de soi. Notre groupe a été, historiquement, l'allié de ces petits indépendants, artisans, commerçants, qui s'appuient sur leurs ressources individuelles pour mener à bien leurs activités et les faire fructifier-

En conclusion, si ce texte n'apparaît pas toujours à la hauteur des enjeux qu'il soulève, se limitant à des considérations trop techniques- il est vrai que d'autres mesures du plan de soutien aux indépendants sont contenues dans le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui un projet de loi dont l'importance et l'actualité doivent être soulignées. La loi Pacte de 2019 se proposait déjà de favoriser la croissance des entreprises à toutes toutes les étapes de leur développement. Sans nier l'intérêt ni l'importance de cette question, notre groupe s'était opposé à l'adoption du projet de loi Pacte, le considérant comme mal ficelé et fourre-tout.

en complément d'une activité salariée. Il y a là un phénomène de société que le législateur doit prendre en compte, mais aussi encadrer, de telle sorte qu'il ne soit pas l'alibi, voire l'aubaine, pour des formes d'emploi dégradées et précaires, comme cela arrive C'est donc avec rigueur et sérieux que nous avons abordé l'examen de ce projet de loi. Et je dois dire d'emblée, pour le regretter, que ni le texte lui-même ni la procédure arrêtée pour l'examiner ne sont complètement à la hauteur d'un tel sujet. Le projet de loi tel qu'il nous est présenté ne répond pas suffisamment à l'objectif de protection. Il ne règle pas le problème de la transmission. Il a été établi avec trop de précipitation.

Nous entamons donc le présent débat parlementaire avec de fortes réserves, qui ne sont toutefois pas des oppositions de principe. Nous souhaitons que ce projet de loi soit sensiblement amélioré afin qu'il protège mieux les entrepreneurs individuels. individuels. Face au faible succès du régime de l'EIRL, le projet de loi tend à en élargir les dispositions à l'ensemble des entreprises individuelles en le simplifiant à l'extrême, et ce sans aucune obligation d'informer les créanciers quant à la consistance du patrimoine professionnel. Dans son avis et dans sa sagesse, le Conseil d'État laisse entendre qu'il était possible de procéder autrement, en améliorant le statut d'EIRL l'allégement des formalités qui lui sont liées et en le faisant connaître plus largement. plus largement. Ce qui nous importe, à nous, c'est la réelle protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur. De ce point de vue, il nous semble qu'il y a un décalage entre l'effet d'annonce et la réalité,

induit- c'est un vrai regret -un amoindrissement de la protection des créanciers du fait du déficit d'information quant à la consistance du patrimoine professionnel de ces entreprises individuelles nouvelle version. nous attacherons donc, par nos amendements, à assurer une protection plus complète du patrimoine personnel de l'entrepreneur et une meilleure information des créanciers.

Vous représentez le fil rouge de mon engagement ces dernières années, le mérite, le travail, la prise de risque et la volonté de transmettre ! » Cette déclaration, qui aurait pu être la mienne tant j'adhère à son contenu, a en réalité été prononcée par le Président de la République voilà dix jours, à la Mutualité, alors qu'il présentait un plan d'aide en faveur des travailleurs indépendants. indépendants sont au coeur de l'action du Gouvernement. Il n'y en a jamais eu autant : la France en compte actuellement près de 3 millions. Le travail indépendant a connu, ces dernières années, un nouveau dynamisme,

Artisans, commerçants, professions libérales, dirigeants de TPE-PME, tous nous font vivre au quotidien. Ils répondent aux demandes de services de proximité et assurent le maintien d'un lien économique et social indispensable dans nos territoires. Ils incarnent des valeurs essentielles pour la vitalité de notre pays : le travail, le sens de l'engagement et de l'effort, l'esprit d'entreprise, le goût pour l'innovation et la transmission des savoir-faire. Le Gouvernement s'est tenu à leurs côtés pendant la crise, grâce notamment à l'ensemble de nos dispositifs de soutien. Mais, comme l'a annoncé le Président de la République le 16 septembre dernier, lors de sa présentation du plan Indépendants, nous devons aller encore plus loin dans l'accompagnement. Ce plan, le premier élaboré depuis vingt-sept ans à l'intention de tous les travailleurs indépendants, comprend une vingtaine de mesures organisées autour de trois exigences d'abord, mieux protéger les indépendants face aux accidents de la vie ; ensuite, mieux accompagner la création d'entreprise et la transmission ; enfin, simplifier les démarches au quotidien.

de renforcer la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur tout en décomplexifiant l'accès à une telle protection, d'une part, et de mettre en extinction le statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée,

la procédure disciplinaire relative aux experts-comptables, ainsi que les règles régissant la gestion des personnels des chambres de commerce et d'industrie. Ce projet de loi peut nous rassembler, je le crois, sur un certain nombre de points

vise tout d'abord à la création d'un statut unique, protecteur du patrimoine personnel, pour l'exercice en nom propre d'une activité professionnelle. Désormais, seuls les éléments utiles à l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel pourront être appréhendés en cas de défaillance. Par cette protection automatique, il sera mis fin aux risques pesant sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel lorsque surviennent des difficultés professionnelles. Il permet, ensuite, de faciliter la transformation d'une entreprise individuelle en société. Le statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée sera mis en extinction progressive, ses principaux avantages étant repris dans le nouveau statut d'entrepreneur individuel. Le texte tend, par ailleurs, à faciliter le rebond des travailleurs indépendants en leur permettant de devenir éligibles à l'ATI, l'allocation des travailleurs indépendants, lorsqu'ils cessent leur activité devenue économiquement non viable. Un décret viendra compléter la réforme de l'ATI par l'assouplissement du critère de revenus de 10 000 euros, qui ne sera désormais exigé que sur la meilleure des deux années. Enfin, nous allons simplifier l'environnement juridique et l'accès des entrepreneurs à l'information

Nous avons essayé de prendre en compte la totalité des étapes de la vie d'un entrepreneur. C'est pourquoi le groupe RDPI votera en faveur de ce texte. La parole

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'accès à l'assurance chômage « pour tous les travailleurs » était une promesse de campagne du futur Président de la République en 2017, les travailleurs indépendants ne disposant pas, à la différence des salariés, d'une protection obligatoire contre le risque de perte d'emploi et n'ayant donc accès qu'aux minima sociaux ou à des assurances privées peu attractives. Le degré d'exposition des travailleurs indépendants au risque de perte d'emploi est inégal. Si, traditionnellement, les indépendants le géraient par eux-mêmes, ce risque peut néanmoins être significatif pour une partie d'entre eux, ce qui provoque une demande de protection justifiant une réforme. La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a donc ouvert des droits au chômage pour les indépendants, avec la création de l'ATI, entrée en vigueur le 1 novembre 2019. Elle a aussi opéré, à bas bruit, un changement profond de la nature de l'assurance chômage en ouvrant la voie à la suppression des contributions salariales et en leur substituant un financement par l'impôt, en l'occurrence par une part de la CSG sur les revenus d'activité.

Lors de l'examen du projet de loi, notre groupe avait souligné le caractère extrêmement restrictif du droit à l'assurance chômage ainsi créé, le texte imposant la réunion de cinq conditions cumulatives que la rapporteure de la commission des affaires sociales, Frédérique Puissat, a rappelées : conditions relatives à la durée d'activité, au niveau de revenus professionnels, aux ressources, à la forme juridique de la cessation d'activité. À sa création, le dispositif de l'ATI visait 29 300 bénéficiaires potentiels, pour un budget de 140 millions d'euros. Le premier bilan apparaît très décevant puisqu'à peine plus d'un millier d'indépendants ont pu bénéficier de cette allocation. Le système retenu s'est révélé complexe et les conditions posées sont apparues Un rapport de l'Assemblée nationale publié en avril dernier sur le sujet évoque une « erreur de ciblage » et souligne que le cumul des cinq conditions qui encadrent l'octroi de l'ATI entraîne incontestablement l'inéligibilité de milliers d'indépendants demandeurs d'emploi. ce rapport parlementaire ont procédé à l'analyse des dossiers traités par Pôle emploi afin d'apporter un début d'éclairage sur les points de blocage. Ainsi, le premier motif de rejet des demandes d'ATI a trait au seuil de revenu minimal d'activité de 10 000 euros annuels, ce critère représentant à lui seul les trois quarts des refus. Par ailleurs, l'exigence d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires exclut de fait un certain nombre d'indépendants, notamment les microentrepreneurs. Aussi le plan de soutien aux indépendants annoncé le 16 septembre dernier par le Gouvernement a-t-il prévu plusieurs aménagements du dispositif de l'ATI, qui figurent en partie dans le présent projet de loi. Il s'agit d'élargir le bénéfice de l'ATI aux cas de « déclaration de cessation totale et définitive d'activité lorsque cette activité n'est pas économiquement viable », ce qui permet de sortir des seuls cas de liquidation ou de redressement judiciaires. Le Gouvernement prévoit également la publication d'un décret assouplissant le critère de revenus de 10 000 euros, qui ne sera désormais exigé que sur la meilleure des deux années. Le Président de la République reconnaissait en effet, lors de la présentation du plan, que la dernière année, qui était systématiquement prise en compte, était rarement la meilleure ... Ces mesures suffiront-elles pour assurer un rééquilibrage de l'ATI ? Disposons-nous de suffisamment de recul pour considérer cette allocation comme un outil utile et viable ? Afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs, d'ici cinq ans d'apprécier la portée de ces ajustements, qui feront l'objet d'une concertation avec les partenaires sociaux. La commission a également prévu une information obligatoire des travailleurs indépendants sur la possibilité de souscrire une assurance contre la perte d'emploi subie. Selon l'association dirigeants sur dix n'auraient jamais entendu parler de cette solution. Il me semblerait d'ailleurs utile, monsieur le ministre, d'améliorer la diffusion de l'information sur l'ATI elle-même, car, en la matière, la méconnaissance peut en partie expliquer le non-recours.

Certes, les travailleurs indépendants ne contribuent pas à l'assurance chômage, mais la substitution croissante de la CSG aux cotisations sociales et les allégements sur les bas salaires modifient l'effort contributif des uns et des autres, sans réflexion sur l'effet de cette modification quant à l'équité entre salariés et non-salariés.

le présent texte en faveur de l'activité professionnelle indépendante comporte des avancées intéressantes. Je pense à la création d'un statut unique, protecteur du patrimoine personnel, pour l'exercice en nom propre d'une activité professionnelle ou à la simplification qu'induit l'extinction progressive du statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Je me suis plus particulièrement intéressée aux articles 9 et 10, délégués au fond à la commission des affaires sociales.

que le régime de la microentreprise, qui a été appelé en 2009 « autoentreprise », n'est pas un statut juridique, mais un régime fiscal et social dérogatoire du droit commun. Ceux qui l'utilisent sont, juridiquement parlant, travailleurs indépendants. Vous précisiez que, à ce titre, ils bénéficiaient des mesures du plan de soutien aux indépendants. Nous savons bien cependant, monsieur le ministre, que le régime de la microentreprise, parce qu'il est vraiment dérogatoire du droit commun, tend à brouiller la compréhension que l'on peut avoir des conséquences qui accompagnent le fait de l'investir et de devenir autoentrepreneur.

De fait, nous pouvons craindre qu'une part considérable d'entre eux ne soient victimes d'un redoutable miroir aux alouettes les conduisant à endosser ce statut et à s'abîmer dans une activité professionnelle relevant des nouvelles formes du travail sans être suffisamment armés et protégés pour cela. Pour mémoire, l'Insee a mis en évidence cette année le fait qu'en 2020 le nombre total de créations d'entreprises avait atteint en France un nouveau record : 848 200 créations soit 4 % de plus qu'en 2019, et ce malgré la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19. Il apparaît ainsi que cette hausse est de nouveau portée par les immatriculations d'entreprises individuelles sous le régime de la microentreprise, en augmentation de 9 %, tandis que les créations d'entreprises individuelles classiques diminuent de 13 %. Dans le même temps, il existe une grande diversité de situations : toujours selon l'Insee, dans l'industrie et le commerce, la médiane des revenus ne dépasse pas 150 euros par mois en 2017, alors qu'elle atteint 500 euros par mois dans la construction. Un quart des microentrepreneurs gagnent plus de 1 000 euros par mois dans les activités immobilières, le conseil de gestion, l'architecture et l'ingénierie. Les nouvelles formes de travail sont nombreuses et protéiformes ; de surcroît, elles changent elles-mêmes rapidement. Elles mettent au défi notre protection sociale, aujourd'hui impuissante à protéger ces nouveaux travailleurs. Je constate que, dans votre projet de loi, il n'y a pas un seul article concernant un certain type d'autoentrepreneurs : les Uber, les Deliveroo et autres « cyberprécaires » des plateformes de travail. Pourquoi n'y sont-ils donc pas mentionnés, malgré l'importance de l'enjeu que représente l'apparition de ces nouveaux modes de travail pour notre économie et pour notre société ? Est-ce parce que votre gouvernement reconnaît, monsieur le ministre, comme le fait la Cour de cassation avant lui, que ces travailleurs sont des indépendants fictifs, et qu'à ce titre leur place est dans le code du travail ?

Face à la complexité des mutations du travail que nous semblons encore incapables d'appréhender, confrontés à la rapidité de leur évolution, on ne se défait pas de l'impression que nous courons après un train lancé en trombe sans parvenir à le rattraper.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, près de 3,2 millions de travailleurs indépendants exercent actuellement en France, couvrant de nombreux secteurs de notre vie quotidienne artisans, commerçants, professions libérales, travailleurs des plateformes, entrepreneurs agricoles ... Tous créent de la richesse, font vivre nos territoires, souvent sans compter leur temps et pour des revenus modestes. L'entrepreneuriat est en France très dynamique ; les créations d'entreprises individuelles ne fléchissent pas, au contraire : on décompte plus de 630 000 créations en 2020. Pourtant, ces dernières années, les indépendants ont dû faire face à plusieurs crises dont l'impact sur leurs revenus a été considérable : crise des « gilets jaunes », grèves contre la réforme des retraites, crise sanitaire. Les secteurs de l'hôtellerie-restauration et de l'événementiel ont particulièrement souffert. Il faut ainsi attendre la fin du quinquennat pour que le Gouvernement annonce un plan spécifique, après quatre années pendant lesquelles les indépendants ont fait l'objet d'une attention toute relative. La mesure principale de ce projet de loi est la mise en place d'un statut unique de l'entrepreneur individuel et la séparation du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel. Il s'agit d'éviter les situations où, ayant choisi le statut d'entrepreneur individuel, l'indépendant doit accepter de voir ses dettes professionnelles recouvrées sur son patrimoine personnel.

Ce nouveau statut simplifiera également la transmission du patrimoine de l'entrepreneur individuel vers une autre entreprise ou vers l'un de ses héritiers, ce qui est positif. Le statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, qui offre plus de garanties, n'a pas été un grand succès. Quelques dizaines d'entreprises seulement sont ainsi créées chaque année- la complexité administrative et les difficultés de financement sont en cause. Ce statut sera donc mis en extinction.

La définition du patrimoine professionnel, qui est assez floue, n'est-elle pas source de contentieux avec les créanciers ? Aussi louable soit ce texte, nous sommes en droit de nous demander s'il est réaliste. Le Gouvernement doit apporter des précisions sur ces points et nous faire part des discussions qu'il mène avec les banques. Un dernier point, sur le cas particulier des artisans : le projet de loi prévoit une habilitation à légiférer par ordonnance pour clarifier le code de l'artisanat.

Herzog, sur l'article. Monsieur le ministre, mes chers collègues, le chapitre I du projet de loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante concerne les différents statuts des entrepreneurs. Le projet de loi vise à les simplifier. Toutefois, il n'aborde pas le statut des conjoints des travailleurs indépendants. Les conjoints sont considérés comme des travailleurs indépendants s'ils participent de manière régulière à l'activité de l'entreprise et sont mariés ou liés par un pacte civil de solidarité au détenteur de l'entreprise individuelle. Ce statut prévoit, pour les entreprises, des cotisations minimales d'environ 30 % ; il représente un intérêt social et fiscal pour la jeune entreprise. Le Gouvernement souhaite modifier ce statut pour limiter la situation de dépendance économique du conjoint à l'égard de l'entreprise et du chef d'entreprise. C'est la raison pour laquelle le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale visera à le supprimer. Ce statut constituait un avantage certain pour l'entreprise, tant pour le chef d'entreprise que pour son conjoint, car il supprimait le travail dissimulé si répandu dans notre pays depuis des décennies. En visant à réduire les situations de dépendance, cette nouvelle mesure va créer de nouveaux problèmes : ce projet de loi n'en parle pas. C'est d'autant plus étonnant que l'on y aborde le problème du patrimoine. Or le patrimoine concerne le couple. Quant au statut d'associé, comment l'appliquer si le conjoint n'exerce pas le même métier ou s'il n'est pas diplômé ? Par exemple, un conjoint non-dentiste peut-il être associé dans un cabinet dentaire et une secrétaire qui n'est pas expert-comptable peut-elle être associée dans un cabinet d'expertise comptable ?

précise des biens qu'ils affectent à leur patrimoine professionnel. Cette simplification à l'extrême des démarches dites « administratives » ne nous paraît par opportune, car elle risque de déséquilibrer le nécessaire lien de confiance et la transparence qui transparence qui conditionnent l'activité économique. Le fait de ne pas être informé sur le patrimoine ne favorise pas la confiance entre les acteurs économiques. Le déficit d'informations sur la consistance du droit de gage donc s'avérer contre-productif, devenir une source d'insécurité et entraver les relations entre professionnels. Cet amendement vise à inciter l'entrepreneur individuel à mettre à disposition de ses créanciers ou fournisseurs une attestation simplifiée et mise à jour chaque année relative à la composition de son patrimoine professionnel. Quel l'avis de la commission ? Mme Blatrix Contat et ses collègues soulèvent une question importante. Dans le régime actuel de l'EIRL, la consistance du patrimoine affecté d'un entrepreneur est connue de tous, notamment de ses créanciers, puisque la déclaration d'affectation doit être accompagnée d'un inventaire des biens affectés. Estimant cette procédure trop complexe, le Gouvernement propose que les entrepreneurs disposent désormais de plein droit de deux patrimoines, l'un professionnel, l'autre personnel, la démarcation entre les deux patrimoines résultant d'un critère légal. À l'évidence, cette réforme, quels qu'en soient les mérites, sera une source d'incertitude pour toutes les personnes en relation d'affaires avec l'entrepreneur individuel, notamment pour ses créanciers. pour ses créanciers. Il est indispensable de veiller à ce qu'elle n'assèche pas complètement le crédit des entrepreneurs individuels. À cet effet, nos collègues proposent que l'entrepreneur individuel soit tenu de mettre à disposition de ses créanciers une attestation, mise à jour annuellement, définissant la composition de son patrimoine professionnel. Le problème, c'est que l'amendement ne précise pas quels seraient les effets juridiques de cette attestation ni les sanctions liées à l'absence d'attestation ou de mise à jour. Faut-il comprendre que l'attestation aurait une fonction constitutive, autrement dit que le patrimoine professionnel serait constitué des éléments figurant dans l'attestation ? On comprend mal comment cela pourrait se concilier avec la définition légale du patrimoine professionnel. En outre, cela reviendrait à maintenir un régime très proche du régime actuel de l'EIRL. L'attestation aurait-elle seulement une fonction probatoire, c'est-à-dire que l'entrepreneur individuel ne pourrait plus contester l'appartenance à son patrimoine professionnel d'un élément figurant dans l'attestation ? Pourquoi pas, mais la commission a institué d'autres règles de preuve qui s'articulent mal avec celle-ci. En outre, cette fonction probatoire de l'attestation impliquerait qu'elle soit publiée et qu'elle ne puisse pas être modifiée à tout moment au gré d'éventuels contentieux, ce que l'amendement ne tend pas à prévoir. Dans ces conditions, il me paraîtrait plus raisonnable de retirer

Afin de dissiper des craintes mal fondées, le présent amendement vise à rattacher expressément au patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel les dettes fiscales dont il pourrait être redevable au titre d'impositions assises sur des biens compris dans son patrimoine professionnel, par exemple la taxe foncière sur les propriétés bâties, assise sur un immeuble compris dans le patrimoine professionnel. Quel est l'avis du

à savoir le fait que cette dette soit née ou non à l'occasion de l'exercice professionnel. Ce critère nous paraît suffisant pour permettre la détermination de la nature professionnelle ou personnelle de chaque type de dette.

de l'entrepreneur individuel pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dus par celui-ci ou par son foyer fiscal, et non pas seulement les biens compris dans le patrimoine personnel, dès lors que l'assiette de ces impositions comprend des revenus tirés de l'activité professionnelle professionnelle de l'entrepreneur. Cette faculté ne pourrait donc s'exercer dans le cas où l'entrepreneur individuel aurait opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés des résultats de son activité professionnelle, comme le prévoit l'article 4 du projet de loi de finances pour 2022.

l'article 1 tendait à prévoir que l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale bénéficient d'une dérogation au principe de séparation des patrimoines. C'était le cas en matière de fraude ou d'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales et sociales, mais aussi pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux, ainsi que de la taxe foncière afférente aux biens immeubles utiles à l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel en ce qui concerne l'administration fiscale. C'était également le cas pour le recouvrement de la contribution sociale sur les

étaient protégées par des dispositions spécifiques qui maintiennent leur droit de gage sur l'ensemble des patrimoines, personnel et professionnel. Il s'agit donc bien d'une protection en faveur des créanciers publics. Or cette inopposabilité a été supprimée en commission des lois au motif qu'elle n'avait pas lieu d'être, sans que soient apportés des éléments explicatifs. comme le souligne le Conseil d'État, ces prérogatives répondent à l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude ainsi qu'à l'objectif d'intérêt général d'effectivité du recouvrement des prélèvements obligatoires en cause. C'est pourquoi il nous semble au contraire important de préserver cette dérogation. Quel est l'avis de la commission

Pour le dire simplement, ce nouveau statut ne changerait rien aux règles de la communauté conjugale, qu'il s'agisse des pouvoirs reconnus aux époux pour administrer les biens communs ou en disposer, ou du sort des dettes nées pendant le mariage. Cette précision est indispensable pour garantir la sécurité juridique de la réforme. À défaut, il risquerait d'y avoir un conflit entre les règles applicables au patrimoine professionnel et celles qui concernent les biens communs éventuellement compris

Le modèle proposé par le Gouvernement, qui sera précisé au niveau réglementaire, est de permettre, avec l'autorisation du conjoint, l'inclusion de biens dans le patrimoine professionnel. Dès lors que ces biens sont dans le patrimoine professionnel, ils ne sauraient être saisis par les créanciers du conjoint. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

Contat. Cet amendement vise à rendre effective la protection du patrimoine de l'entrepreneur, plus particulièrement particulièrement de sa résidence principale. Les conséquences d'une cessation d'activité d'un travailleur indépendant peuvent être extrêmement graves socialement et familialement si elles vont jusqu'à la confiscation du logement familial. 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a mis en place une protection par défaut, sans déclaration d'insaisissabilité devant notaire. Cette mesure a permis de répondre à la question du déficit d'information

n'a pas pour effet de remettre en cause l'insaisissabilité de sa résidence principale, qui résulte de l'article L. 526-1 du code de commerce. est pleinement satisfait par le texte de la commission, qui dispose, en son alinéa 18, que le nouveau statut de l'entrepreneur individuel doit s'entendre sans préjudice des dispositions légales relatives, notamment, à l'insaisissabilité de biens immobiliers. Je demande donc le retrait de cet amendement.

d'indépendants. Des sociétés de caution mutuelle structurées et dédiées existent pour assumer ce type de risque, tant pour les artisans que pour les commerçants ou les professionnels libéraux. Cette solution n'est toutefois pas proposée systématiquement à ce jour par les conseillers bancaires. Cet amendement vise donc à rendre systématique la proposition d'une alternative sous forme de garantie par une société de caution mutuelle. Mme Berthet et ses collègues proposent qu'un entrepreneur individuel ne puisse renoncer à la séparation de ses patrimoines au bénéfice d'un établissement de crédit que si celui-ci lui a préalablement « proposé » une « offre de garantie par une société de caution mutuelle », et qu'il l'a refusée. L'intention est tout à fait légitime. Il faut encourager le recours à ces mécanismes de garantie mutualisés plutôt que d'exiger systématiquement des garanties personnelles de l'emprunteur. Néanmoins, le dispositif présenté ne fonctionne pas. On ne peut pas imposer à une banque de proposer à l'un de ses clients une offre de contrat avec une personne tierce. Plus précisément, le recours à une société de caution mutuelle fait intervenir plusieurs contrats : un contrat de société par lequel l'emprunteur devient associé de la société de caution mutuelle, contrat auquel la banque n'est pas partie ; et un contrat de cautionnement entre la société de caution mutuelle et la banque, auquel l'emprunteur n'est pas partie. En pratique, même si l'emprunteur et la banque étaient d'accord, rien n'obligerait la société de caution mutuelle à admettre l'emprunteur parmi ses membres ni à garantir son emprunt. C'est la raison pour laquelle je demande

sens, doivent davantage être protégés face à des aléas économiques parfois mal anticipés. Une telle protection nécessite un diagnostic éclairé sur les perspectives économiques de leurs entreprises. Le présent amendement vise simplement à ce que la création de l'entreprise individuelle soit conditionnée à la réalisation préalable d'une étude de marché qui démontrerait sa viabilité économique. Le porteur du projet pourra donc s'appuyer sur l'expertise des chambres de commerce, des universités ou des organismes de formation.

amendement fait suite aux discussions entre le rapporteur et le Gouvernement depuis l'examen du projet de loi en commission. Dans le cas où le patrimoine professionnel transféré à titre universel comprendrait des dettes pour le recouvrement desquelles la séparation des patrimoines n'était pas opposable aux créanciers, du fait d'une renonciation, par exemple, il est légitime non seulement que l'auteur du transfert reste solidairement obligé à la dette, mais qu'il y contribue également. Il convient donc de fixer par la loi non seulement le principe de co-obligation solidaire, mais aussi celui de la contribution respective de l'auteur et du bénéficiaire du transfert. Or il est conforme à la logique des diverses exceptions au principe de séparation des patrimoines, notamment de la renonciation, que l'auteur du transfert ne contribue à la dette que pour le montant de celle-ci qui excède la valeur des biens et droits compris dans le patrimoine professionnel transféré. En pratique, les créanciers concernés pourraient obtenir de l'auteur comme du bénéficiaire du transfert le paiement intégral de leur créance. Dans le cas où il aurait payé, l'auteur du transfert pourrait se retourner contre le bénéficiaire pour se faire rembourser, dans la limite de la valeur des biens et droits compris dans le patrimoine professionnel transféré.

l'entrepreneur indépendant cédant et le bénéficiaire peuvent rester solidaires envers certains créanciers. Ils déterminent amiablement leur contribution respective à la dette, mais, à défaut, ils peuvent être tenus chacun par moitié.

? Nos collègues proposent que le bénéficiaire du transfert doive être obligatoirement informé de l'existence et de la consistance de telles dettes. Cela ne me paraît pas nécessaire, car il s'agit bien de dettes professionnelles qui, par principe, lui sont cédées. En outre, le fait que l'auteur du transfert reste obligé à la dette et y contribue est protecteur pour le bénéficiaire du transfert. Enfin, l'amendement ne précise pas quelle serait la sanction si l'auteur du transfert manquait à son obligation d'information. Je demande donc le retrait de l'amendement n° 18 rectifié au profit de

tel cas le droit de préemption des coïndivisaires ainsi que le droit de retrait litigieux.

en effet payer des cotisations sociales sur la plus-value lors de la vente du patrimoine bâti professionnel. S'il était en société, il serait simplement assujetti

de décès, « l'entrepreneur n'est pas assujetti aux cotisations sociales sur le patrimoine bâti professionnel intégré au patrimoine personnel ». J'ai quelque difficulté à comprendre le dispositif proposé, car les cotisations sociales ne sont pas assises sur des biens immobiliers, mais sont assises

L'article L. 145-16 du code de commerce répute non écrites les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail commercial ou les droits afférents « à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise ». La notion d'entreprise étant mal définie en droit, il est proposé, pour lever toute ambiguïté, d'étendre expressément cette règle au cas de transfert universel du patrimoine professionnel. Quel est l'avis du Gouvernement ? Il est

rapporteur. Les contrats de travail compris dans le patrimoine professionnel d'un entrepreneur individuel subsisteront de plein droit entre le personnel et le nouvel employeur en cas de transfert universel du patrimoine professionnel. Cet amendement vise à dissiper toute interrogation à ce sujet. Quel est l'avis

ou de redressement est très pénalisante. Cette interdiction peut durer plus d'un an, ce qui rend d'autant plus compliquée la vie de l'entreprise déjà en difficulté. La levée de cette interdiction n'intervient qu'en cas d'homologation d'un d'arrêt des plans ou des jugements de clôture ou de redressement, ou de procédure de rétablissement professionnel. Le présent amendement vise à permettre également cette levée d'interdiction bancaire dès la constatation d'une conciliation amiable. Pour les Pour les entrepreneurs individuels en difficulté, la modalité supplémentaire de levée d'interdiction ainsi créée s'appliquerait aux comptes afférents au patrimoine visé par la procédure. Quel

pour recouvrer cette faculté, de justifier qu'il a réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante. À défaut, et si l'entreprise est par la suite soumise à une procédure amiable de traitement des difficultés ou à une procédure collective, l'interdiction d'émettre des chèques continue évidemment de produire ses effets. En revanche, lors de la clôture de la procédure, si l'entreprise n'est pas liquidée, le chef d'entreprise retrouve la faculté d'émettre des chèques. Cela suppose qu'un tribunal se soit prononcé, qu'il ait constaté la viabilité de l'entreprise et vérifié que les intérêts des créanciers sont correctement pris en compte. Ainsi, la mesure d'interdiction cesse de plein droit de produire ses effets soit lors du jugement d'homologation d'un accord de conciliation, soit lors du jugement arrêtant un plan de sauvegarde ou de redressement. Mme Vermeillet souhaiterait que la mesure d'interdiction d'émettre des chèques cesse également de produire ses effets en cas d'accord de conciliation simplement constaté, et non homologué,

Le tribunal doit notamment vérifier que l'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. Or parmi ces créanciers peuvent également figurer des entreprises ou des entrepreneurs eux-mêmes susceptibles de connaître un défaut de paiement en raison du rejet d'un chèque sans provision.

L'objet de cet amendement est de favoriser la dématérialisation des procédures administratives auxquelles sont soumis les travailleurs et entrepreneurs indépendants lors de leurs différentes démarches. La loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, dite loi Essoc, consacre un chapitre à la dématérialisation des relations entre les usagers et l'administration- les articles 40 à 48 -où s'exprime le principe du « dites-le-nous une fois ». La dématérialisation figure aussi dans la stratégie nationale d'orientation de l'action publique annexée à cette loi. La loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique comporte, elle aussi, des dispositions dans ce domaine. Toutefois, les procédures concernant les travailleurs et entrepreneurs indépendants apparaissent encore souvent trop lourdes et insuffisamment à jour au regard des moyens de communication actuelle. Certaines difficultés se sont d'ailleurs révélées tout particulièrement durant la pandémie. dans ma question écrite du 17 décembre 2020, ai-je interrogé le Gouvernement sur la dématérialisation de la procédure fiscale des droits d'enregistrement par la direction générale des finances publiques. Il est ici proposé de demander un rapport au Gouvernement sur ces expérimentations, sans se limiter aux seules questions fiscales, pour toucher le plus large éventail possible de procédures concernant les indépendants. Quel est l'avis de la

son patrimoine affecté à une autre personne, l'affectation serait maintenue de plein droit, avec pour conséquence la soumission du bénéficiaire du transfert au régime de l'EIRL s'il n'y était pas déjà soumis.

de s'y soumettre à l'avenir, il est en revanche légitime qu'un EIRL puisse céder l'un de ses patrimoines affectés à un autre EIRL existant, avec maintien de l'affectation.

ce projet de loi. Cet article habilitait le Gouvernement à prendre une ordonnance afin de simplifier l'exercice en société des professions libérales réglementées. Tout d'abord, je tiens à souligner que cette réforme a fait l'objet d'un travail approfondi et d'une première phase de concertation avec les organisations professionnelles à la suite de la remise du rapport de l'inspection générale des finances en novembre 2020. Il y a 68 organisations professionnelles dans les professions libérales ;

le premier constat est partagé entre nous : l'exercice sous forme sociétaire des professions libérales réglementées, s'il demeure minoritaire- environ les deux tiers des professionnels libéraux exercent en tant qu'indépendants -répond à un réel besoin de ces professionnels, leur permettant de mutualiser des moyens, d'anticiper le développement de leur activité, ou tout simplement de s'inscrire dans une perspective de long terme et de transmission. C'est la raison pour laquelle ce sujet important trouve une place naturelle dans le cadre du projet de loi que je porte. Le second constat est tout aussi consensuel : cet exercice en société demeure aujourd'hui complexe, parfois même dissuasif. C'est notamment le résultat de la superposition et de l'enchevêtrement, pour reprendre les termes de votre rapporteur, de textes juridiques nombreux. Cet état de fait est source d'incertitude et d'insécurité juridique pour les professionnels libéraux. La nécessité de légiférer est, à ce titre, établie sans conteste. Sur la base de ces constats, je retiens deux réserves exprimées par la commission. Premièrement, les problématiques propres aux différentes professions seraient trop diverses pour permettre de les traiter ensemble. Deuxièmement, la question de l'ouverture du capital serait trop sensible et susciterait trop d'interrogations. Je reviendrai tout d'abord sur ce dernier point. Nous ne prendrons dans cette ordonnance aucune initiative qui ne soit pleinement consensuelle avec les professionnels concernés. le répète : nous ne prendrons aucune initiative qui ne soit pleinement consensuelle avec les professionnels concernés. Ainsi, toutes les écritures qui trouveront place dans l'ordonnance seront coconstruites avec eux en amont et soumises à concertation en aval. Il en va ainsi, bien évidemment, de la question sensible de l'ouverture du capital. Je me permets d'ailleurs de préciser que cet axe de nos travaux couvre également la question de l'assouplissement du régime des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL), qui fait l'objet d'un large consensus. L'autre réserve tenait à la diversité des situations rencontrées et des souhaits potentiellement divergents qui peuvent se manifester au sein des différentes familles de professions libérales. Sur ce point, je rappellerai tout d'abord que les textes en vigueur, en particulier la loi du 31 décembre 1990 sur les sociétés d'exercice libéral, comportent déjà des dispositions visant spécifiquement telle ou telle famille professionnelle. Notre objectif est très simple : nous souhaitons clarifier les règles applicables aux professions libérales, tout en opérant une distinction précise entre ce qui relève d'un socle commun à l'ensemble de ces professions et ce qui est et restera propre à chaque famille. C'est en cela que le vecteur de l'ordonnance nous paraît incontournable, au regard du nombre et de la technicité des textes à rationaliser ou à rapprocher, y compris à droit constant. une fois cette difficulté résolue, notre approche aura l'immense avantage de mettre en regard les dispositions comparables qui s'appliquent aux uns et aux autres, en y intégrant des problématiques éminemment interprofessionnelles, comme le développement des sociétés pluriprofessionnelles d'exercice, dont le statut demeure largement perfectible. Permettez-moi aussi de vous préciser que nous allons entrer dans une seconde phase de consultation approfondie, qui va permettre de creuser les sujets déjà identifiés et sûrement d'en faire apparaître d'autres.

J'ai bien entendu également le souhait du Sénat d'être associé à ces travaux. Je vous propose que des concertations dédiées puissent être menées avec vos représentants afin de recueillir leurs contributions sur ces sujets sensibles et de les ajouter à celles que nous obtiendrons directement auprès des professionnels.

du 31 décembre 1990 plafonne les comptes d'associés à hauteur de trois fois leur participation au capital : M. Y et Mme Z ne peuvent donc pas avancer les fonds nécessaires à leur investissement. Après la réforme, les comptes d'associés sont déplafonnés : M. Y et Mme Z peuvent compléter leur trésorerie sans recourir à un prêt bancaire. exemple est celui de M. K, radiologue : il exerce au sein d'une société d'exercice libérale et souhaiterait devenir propriétaire de ses locaux. Il a créé une société holding pour structurer ses investissements au sein de sa société.

habilitait le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour préciser les règles communes applicables aux professions libérales réglementées et adapter les différents régimes d'exercice sociétaire. L'habilitation visait également à faciliter le développement et le financement des structures d'exercice de ces professions. À partir de là, nous allons diverger, je le crois ... Je le crains ... Commençons par le fond. La superposition de régimes juridiques permettant l'exercice sociétaire des professions libérales réglementées est certes regrettable et le droit mériterait une clarification. Pour autant, il n'existe pas de consensus au sein de ces professions sur le sens à donner à une telle réforme. Certaines sont opposées tant à la convergence des régimes d'exercice sociétaire qu'à la modification des règles relatives à la détention du capital et à la répartition des droits de vote. D'autres professions sont favorables à ces deux points et certaines s'opposent uniquement au second. Les modifications relatives aux règles de détention du capital et de répartition des votes suscitent, de mon point de vue, les plus fortes interrogations. Il est en effet crucial de préserver les garanties d'indépendance caractérisant l'exercice des professions libérales réglementées.

qu'« aucune modification ne saurait être envisagée, ou aboutir, sans l'appui des professions concernées ». Monsieur le ministre, ne confondons pas vitesse et précipitation ! Vous l'avez déjà fait à plusieurs reprises et vous avez entendu le Sénat à ce sujet.

les concertations menées par le Gouvernement ne sauraient en aucun cas, à notre sens, se substituer à un débat parlementaire. La promesse du Gouvernement de n'agir qu'avec l'appui des professionnels ne peut pas

Depuis une dizaine d'années, le recours aux ordonnances dans des domaines relevant normalement de la loi est devenu plus fréquent ; il s'est même banalisé durant ce quinquennat dans des proportions sans commune mesure avec ce que la V République avait connu jusqu'à présent. Depuis 2017, plus de la moitié des textes relevant du domaine de la loi sont pris par ordonnance. En 2020, on a atteint un record : 73 % des textes sont des ordonnances l'évidence, faire passer une mesure sans recourir au débat parlementaire est devenu une marque de fabrique de cet exécutif ; c'est très révélateur de la posture « jupitérienne » du Président de la République. Rappelons que la force de l'article 38 de la Constitution se trouve dans son utilisation parcimonieuse. En y ayant trop souvent recours, on retire au Parlement sa capacité de faire la loi. Parce que le Parlement ne doit pas être considéré comme une simple chambre d'habilitation et qu'il doit pleinement assumer son rôle et ses compétences, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires demande que les clarifications, la rédaction et le plan du code de l'artisanat soient réalisés par la voie législative.

fixé. Ajoutons-y le fait qu'en raison d'une récente jurisprudence du Conseil constitutionnel certaines ordonnances ne donnent désormais plus lieu à ratification par le Parlement, et l'on ne peut être que prudents à l'égard du recours à cette nouvelle façon de légiférer. Ensuite, il est indiqué, dans ce même article 7, que l'ordonnance pourra également « actualiser les dispositions applicables » aux départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, « en procédant aux adaptations nécessaires

bien sûr interrogée sur l'intérêt de cette demande d'habilitation à légiférer par ordonnance, compte tenu du recours croissant à cette procédure. Certes, nombre de demandes d'habilitation ne sont pas nécessaires, contournent

Je vous rappelle par ailleurs, mes chers collègues, que cet article prévoit que la codification se fera à droit constant, c'est-à-dire sans ajout de dispositions qui n'auraient pas été débattues par nos assemblées.

cet article 7, qui permet au Gouvernement de légiférer par ordonnance sur ce point. Je m'engage naturellement, monsieur le rapporteur pour avis, à ce que ces travaux se fassent en parfaite

Ce rapport m'a été remis il y a quelques semaines, et je recevrai dans quelques semaines les présidents d'exécutifs locaux nouvellement élus dans cette région afin que l'on puisse adapter le fonctionnement de la chambre régionale à la situation particulière de l'Alsace et de la Moselle.

certains délais et certaines procédures s'imposent à l'administration, comme vous venez de le rappeler, sans qu'ils puissent lui être imputés. En effet, l'exercice de codification mêle plusieurs acteurs, dont la commission supérieure de codification, qui n'aura pas à étudier que ce texte.

permanent de celles-ci. Le présent amendement vise à ajouter à ladite liste l'activité de toilettage des chiens, chats et autres animaux de compagnie. Et des défendons la nécessité de subordonner l'installation de toute activité de toilettage, qu'elle s'exerce en salon, de manière itinérante, ou à domicile, à l'obtention, par au moins une personne en contact direct avec les animaux, d'un diplôme ou d'un titre

Le règlement européen dit « loi de santé animale » du 9 mars 2016 est entré en vigueur le 21 avril 2021. Ce texte fixe les modalités de prévention et d'éradication des maladies animales transmissibles et renforce la biosécurité. Les opérateurs- c'est-à-dire les salariés, les chefs d'entreprise, ou les propriétaires de chiens ou chats

La commission considère qu'une telle disposition va dans le bon sens, les manipulations sur animaux pouvant induire des souffrances et des dégâts si elles ne sont pas correctement réalisées. En outre, renforcer la professionnalisation de ces métiers permettra un contrôle accru permettant de détecter d'éventuelles maladies animales.

est ainsi libellé : La parole est à M. Éric Gold. Par cet amendement, nous souhaitons contribuer à mettre un terme aux cautions personnelles des dirigeants indépendants pour les emprunts souscrits à des fins professionnelles. Actuellement, lors de la souscription d'un emprunt professionnel, le dirigeant doit le plus souvent apporter une caution sur ses biens personnels. Cette situation représente un risque financier disproportionné pour les exploitants individuels, souvent confrontés à des difficultés dans leurs projets d'investissement et d'emprunt auprès des banques. Pour encourager l'esprit d'entreprise, il faut que les risques soient équitablement répartis entre les différents acteurs économiques. Or ce projet de loi ne nous semble pas répondre de façon satisfaisante à cette question sensible des cautions personnelles. C'est pourquoi nous proposons dans cet amendement ces cautions dans le mécanisme de garantie des cautions prévue à l'article L. 313-50 du code monétaire et financier. Cela pourrait notamment contribuer à lever les réticences des établissements bancaires à accorder des crédits aux entrepreneurs individuels en l'absence de caution personnelle, ou à limiter les demandes de telles cautions. Quel est l'avis de

doit à tout moment justifier d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement des salaires des intérimaires. Or les banques et autres établissements de crédit qui fournissent ces garanties obligatoires sont eux-mêmes exposés à un risque de défaillance. C'est pourquoi la loi leur impose de contribuer au financement d'un mécanisme de garantie des cautions géré par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution

pour répondre à un problème bien connu, à savoir le fait que les dirigeants de sociétés personnelles à responsabilité limitée sont très souvent appelés à cautionner sur leur patrimoine personnel les emprunts de leur société, ce qui revient à les priver de la protection offerte par la création d'une société. je le reconnais, est éminemment légitime, mais le dispositif est manifestement inconstitutionnel, puisqu'il revient à imposer à un fonds financé par les seuls établissements de crédit de couvrir le risque de défaillance des dirigeants de sociétés unipersonnelles qui se sont portés cautions pour leur société. Il y a là une rupture caractérisée d'égalité devant les charges publiques.

La création de l'ATI s'inscrit dans la dynamique d'harmonisation de la protection sociale des salariés et des indépendants mise en oeuvre au cours des dernières années, qui tend à rapprocher les droits sociaux des travailleurs indépendants de ceux des salariés tout en tenant compte de leurs spécificités professionnelles. La création de l'ATI répond également à l'objectif de les protéger contre le risque de défaillance de leur entreprise. Il s'agit ainsi de sécuriser les transitions professionnelles des indépendants en leur offrant un filet de sécurité leur permette d'être indemnisés le temps de rechercher une nouvelle activité, lorsque leur entreprise cesse la sienne de manière définitive. Elle répond aussi à la nécessité d'adapter le système français de couverture du risque chômage à la diversification accrue des formes de travail et d'emploi, qui remet en cause les frontières entre travail salarié et non salarié.

mesures de ce plan. En théorie, l'ATI est censée couvrir les travailleurs des plateformes, mais les conditions de ressources, de durée d'activité et de revenus antérieurs d'activité, ainsi que le critère de cessation de l'activité du fait d'une liquidation judiciaire ou d'un redressement judiciaire, excluent de fait la grande majorité des travailleurs de plateforme du bénéfice de ce dispositif. Le rapport Frouin a ainsi estimé que seules 751 demandes d'ATI formulées par des travailleurs des plateformes, sur un ont abouti effectivement à une ouverture de droits. Le principal motif de rejet est un revenu annuel minimal d'activité inférieur à 10 000 euros. En outre, environ un tiers des travailleurs potentiellement éligibles ne renvoie pas le questionnaire qui leur a été adressé. Nous estimons donc que l'ATI n'est pas un dispositif adapté à ces travailleurs ; il ne nous paraît pas que les inflexions apportées dans ce projet de loi pourront changer significativement la donne pour eux. C'est pourquoi nous proposons, dans cet amendement, que le bilan de l'ATI prévu en 2024

Certes, le nombre de personnes couvertes est faible, mais cela ne s'explique pas uniquement par la méconnaissance de cette possibilité. Les artisans et les professions indépendantes connaissent bien les assurances ; ils y renoncent pour des raisons financières, en raison de leur coût élevé.

du texte en commission, prévoit une information obligatoire, par des organismes publics, sur la possibilité de recourir à une assurance privée contre la perte de revenu. Cette disposition est présentée comme une réponse à la trop faible utilisation des contrats assurantiels contre le risque de perte d'emploi subie. Elle est, par là même, présentée comme un complément de la facilitation de l'accès à l'allocation des travailleurs indépendants, que prévoit très utilement l'article 9, visant à sécuriser et renforcer la protection de ces non-salariés. L'inscription dans la loi d'une telle obligation d'information peut apparaître discutable, d'autant que la faible couverture peut s'expliquer par d'autres facteurs que le déficit d'information, tels que le coût élevé de certaines assurances par rapport à la nature de l'activité en question. C'est pourquoi, par le présent amendement, nous proposons de ne pas retenir l'article 9 , introduit lors de l'examen du

L'ancien stage de préparation à l'installation répondait bien aux besoins d'accompagnement et de conseil à cet égard. Alors que débutait l'examen de ce projet de loi qui modifie les conditions d'exercice de l'entrepreneur individuel en mettant en oeuvre un nouveau statut, il m'a semblé utile de renouer avec cette ancienne pratique, qui rendait bien des services. Auparavant, c'étaient les chambres de métiers et de l'artisanat qui, en premier rang, organisaient ces stages, qu'elles finançaient au moyen des redevances payées par les stagiaires. À ma connaissance, les recettes recueillies à cette occasion ont toujours permis à tout le moins- c'est presque un euphémisme ! -d'équilibrer ces dépenses. Dès lors, opposer à l'amendement visant à recréer ce stage l'article 40

45 de la Constitution. Les plateformes ont une responsabilité sociale, qui s'exerce par la prise en charge des éventuelles cotisations d'assurance souscrites à titre volontaire par le travailleur contre le risque d'accident du travail. Cette responsabilité induit également une contribution de la plateforme à la formation professionnelle et à la prise en charge des frais d'accompagnement de la validation des acquis de l'expérience. Toutefois, le travailleur ne peut bénéficier de ces prises en charge que s'il a réalisé sur une plateforme un chiffre d'affaires au moins égal à 13 du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 5 268,12 euros en 2019, si bien que ces dispositions semblent concerner peu de travailleurs en pratique. J'attire donc l'attention sur le fait qu'il nous paraîtrait équitable et juste que les plateformes numériques abondent sans condition les comptes personnels de formation des travailleurs auxquels elles font appel et qu'elles veillent à remplir leurs obligations en matière de formation vis-à-vis de ces travailleurs dès que la relation de travail est formalisée. Ainsi, les travailleurs des plateformes seraient un peu moins pénalisés en ce qui concerne l'ouverture de leurs droits à la formation. Que vient faire l'article 45 de la Constitution en la matière ? Je ne comprends pas

en prévoyant que la part dédiée à leur formation professionnelle relève d'un seul fonds d'assurance formation. Il modifie à cette fin les dispositions de l'article L. 6331-48 du code du travail relatif au versement de la contribution à la formation professionnelle des travailleurs indépendants, ainsi que celles des articles relatifs à la répartition de ces fonds par France compétences. Toutefois, les représentants des artisans et des professionnels libéraux s'inquiètent,

Dans ce contexte, le présent amendement vise à inscrire dans la loi que cette répartition doit être effectuée sur le fondement de la nature de l'activité du travailleur indépendant. Quel est l'avis de la commission

le Gouvernement propose, dans le présent amendement, d'exclure de tout mandat exécutif les élus des organismes ayant par ailleurs une activité de formation. Ces élus pourront toutefois participer à tout autre aspect de la vie de ce fonds.

Nous sommes très réservés sur ce choix politique : il est à craindre que l'organisation de nouvelles élections, dans ce climat très tendu et très perturbé, ne permette pas, à elle seule, de sortir de l'impasse. Par ailleurs, l'article 12 contient une série de dispositions de nature à semer le trouble quant aux intentions du Gouvernement sur l'avenir du personnel des CCI

pour le régime de droit privé que l'article 40 de la loi Pacte bornait dans le temps et, d'autre part, en systématisant le principe du remplacement d'éléments statutaires par leur équivalent issu de la convention collective ou d'accords collectifs,

Par ailleurs, il accélère l'extinction du statut d'agent public et des droits afférents, en modifiant l'article L. 712-11 du code de commerce, et il ouvre la voie à l'application de ces nouvelles dispositions conventionnelles aux agents publics.

Premièrement, il n'est pas exact d'affirmer que cet article traduit le choix de ne pas reprendre le dialogue social. En effet, le dialogue est en cours. Seulement, la signature de la convention collective, point d'aboutissement de ce dialogue, n'a pas eu lieu et les salariés de droit privé ne sont donc couverts par aucune convention.

en 2017, lorsque les effectifs des CCI étaient encore tous sous statut de droit public. Il ne me semble pas qu'il faille rejeter cette occasion d'organiser de nouvelles élections, cinq ans après les dernières. Cette démarche saine et positive vise non pas à contourner l'intersyndicale qui représente aujourd'hui les agents sous statut, mais simplement à actualiser la véritable représentativité des syndicats afin que la négociation se fasse entre des organisations reflétant réellement la nouvelle composition des effectifs.

la loi Pacte prévoyait la mise en place au plus tard neuf mois après l'entrée en vigueur de la loi, soit le 29 février 2020. Les difficultés liées à la crise sanitaire nous ont conduits à reporter ce délai au 31 décembre

L'instance représentative nationale du personnel représente les agents publics et les salariés de droit privé des CCI, lesquelles sont restées, je tiens à le rappeler, des établissements publics à caractère administratif. Aussi, il nous paraît nécessaire que l'État reste impliqué dans les relations sociales et le dialogue social au sein des CCI. Sa présence permettrait également à l'État de mieux jouer son rôle de médiation.

Or votre amendement, ma chère collègue, tend à aller plus loin encore : le ministère serait désormais partie prenante de l'instance représentative. Il me semble préférable que les négociations au sein de cette instance aient lieu naturellement entre les parties concernées, c'est-à-dire entre les employeurs que sont les CCI et leur personnel.

il s'agit de veiller au bon usage du produit de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie qui pèse sur les entreprises. Dans cette logique, il nous paraît cohérent que la convention collective s'applique uniquement au personnel de droit privé qui ne bénéficie d'aucun accord pour l'instant. En effet, les salariés employés indirectement sont, pour leur part, déjà couverts par diverses conventions propres à leurs secteurs respectifs. Il paraît contre-productif et lourd pour le réseau de prévoir deux conventions concurrentes pour les mêmes salariés,

Compte tenu de la multitude d'activités gérées indirectement par les CCI, il est tout à fait normal que la convention collective ne soit pas la même pour tous : pour le service de sécurité d'un aéroport, pour les enseignants des écoles de commerce, pour les employés des ports de commerce, pour les conseillers clients, etc. La

loi organise l'extinction programmée du statut des agents publics en systématisant le principe du remplacement d'éléments statutaires par leur équivalent issu de la convention collective.

C'est donc bien le document issu des négociations et du dialogue social qui permettra de prévoir que telle ou telle disposition de la convention remplacera celle du statut, ou qui l'empêchera., ce sont donc bien les organisations syndicales qui gardent la main.

Il s'agit simplement de prévoir une corde de rappel, un filet de sécurité, au cas où le blocage actuel persisterait et où un tiers des effectifs du réseau continuerait à n'être couvert par aucune convention collective. Il s'agit donc bien plutôt d'une mesure bienvenue de protection.

Il importe que de nouvelles élections puissent avoir lieu, les dernières s'étant tenues en 2017. Les représentants actuels bénéficient d'une prolongation de leur mandat, qui ne peut pas être indéfinie.

qui les concerne. Le délai de six mois est suffisant pour négocier un protocole électoral, arrêter le règlement intérieur du CSE et organiser des élections. Une petite accélération devra peut-être être donnée, mais nous sommes confiants dans la capacité du réseau à organiser des

continuent d'être gérées par la commission paritaire nationale existante. L'article 12 prévoit en effet que les CSE seront désormais des organes représentatifs du personnel. est vrai que cette transformation se fait avec, en toile de fond, l'idée que l'ensemble des effectifs sera à terme de droit privé, tandis que la commission paritaire gérait plutôt les agents sous statut.

Par ailleurs, le code de commerce prévoit explicitement que les relations collectives, tant pour les agents de droit public que pour ceux de droit privé, sont régies par le code du travail. Cet amendement est donc déjà satisfait. La commission en demande le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

entre notre rédaction et celle que vous proposez. Premièrement, le Gouvernement souhaite que le régime de l'EIRL soit mis en extinction immédiate, sans attendre l'entrée en vigueur du nouveau statut de l'entrepreneur individuel.

prévu dans le texte de la commission. Un délai de trois mois nous avait paru un peu court pour permettre à l'ensemble des acteurs, notamment aux banques, de s'adapter, mais je veux bien me rallier à cette position. Troisièmement, le Gouvernement souhaite que le nouveau statut impliquant la séparation des patrimoines professionnels et personnels de l'entrepreneur individuel ne s'applique pas aux créances personnelles antérieures à l'entrée en vigueur de la loi. Il me semble qu'il y a là une légère contradiction avec le fait que, pour l'avenir, le Gouvernement prévoit l'application immédiate du nouveau régime aux créances antérieures au commencement de l'activité professionnelle indépendante d'une personne physique. Dans un cas, le Gouvernement considère que l'atteinte aux conventions légalement conclues est disproportionnée ; dans l'autre, qu'elle est proportionnée. Je ne suis pas entièrement

En effet, les chefs d'entreprise artisanale cotisent tant au Fafcea qu'aux conseils régionaux de la formation gérés par les chambres de métiers et de l'artisanat. Les deux organisations disposent du même fichier et le reversement effectué, durant l'année 2022, par le Fafcea aux conseils régionaux de la formation pour la fraction au titre du financement des formations transverses ne poserait aucune difficulté technique. Ensuite, les erreurs d'affectation de la contribution de la formation professionnelle des travailleurs indépendants qui posent problème ne concernent pas la répartition de cette contribution entre le Fafcea et les conseils régionaux de la formation, dont les ressources proviennent des mêmes chefs d'entreprise artisanale, mais sont dues au fait que les contributions d'artisans ou de professionnels libéraux, qui devraient revenir au Fafcea, sont versées de façon erronée à un autre fonds d'assurance formation, à

Il y a pourtant urgence. Notre droit, nous le savons, est devenu inadapté. De nouvelles formes de travail ne sont pas régulées : le dialogue social y est bafoué et les employés y sont mal protégés. Il est grand temps que ce gouvernement assume son inaction, qui est intenable face à la multiplication des situations de salariat déguisé. Cet état de fait est injuste socialement et fragilise notre système de sécurité sociale en entier. Cette inaction est également intenable face aux coups de semonce de la justice. La Cour de cassation a reconnu le statut de salarié aux chauffeurs Uber

et qu'il ne traite pas de l'ensemble des sujets qui intéressent les travailleurs indépendants, notamment leurs relations avec les plateformes. Un texte à ce sujet devrait bientôt être examiné par la commission des affaires sociales. Néanmoins,

3 millions d'entrepreneurs qui, en vertu du principe d'unicité du patrimoine, voyaient leurs patrimoines professionnel et personnel confondus. Ce texte est vraiment

vote. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous achevons l'examen de ce projet de loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante. Il s'agit à nos yeux d'un texte important, puisqu'il aura vocation à s'appliquer à un grand nombre de nos concitoyens. Les modifications apportées par la commission des lois, ainsi que par la commission des affaires sociales et la commission des affaires économiques, étaient nécessaires et attendues. Nécessaires, car la création d'un nouveau statut unique doit constituer une avancée pour les entrepreneurs individuels d'aujourd'hui et de demain. Le groupe Les Républicains se réjouit ainsi de la sécurisation juridique du dispositif effectuée par le rapporteur Attendues, car l'entrepreneuriat individuel connaît un succès chaque année renouvelé et suscite un attrait de plus en plus fort au sein des jeunes générations. Or nous nous devons de les accompagner du mieux possible. Nous nous félicitions également des différentes initiatives des rapporteurs visant à supprimer les habilitations données au Gouvernement à légiférer par ordonnances, notamment celle qui devait lui permettre de réformer ainsi le droit applicable à l'exercice en société des professions libérales réglementées.